et portant diverses dispositions intéressant la défense dans l'édition des articles nous sommes parvenus à l'amendement 124 rectifié au sein du rapport annexé. Et nous commençons par ce fameux amendement 124 qui est défendue par monsieur Perrin.

une interview du ministre des armées, qui avait indiqué en février 2023 à propos des munitions télé-opérées qu'il fallait. Avoir la masse et. Et des objets produits à faible coût. L'objectif est donc d'avoir à terme un stock de 1800 minutes. cet amendement a pour objet d'inscrire dans la LPM, le nombre de munitions télé-opérées donc 1800. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs. Favorable après faut qu'on retienne dans la méthodologie que c'est donc, à titre d'exemple, on donne cet exemple là, mais que d'autres éléments du patch munitions ne figureront pas forcément pour le pour le tableau mais de fait, ça correspond à ce qui est dans la copie, donc avis favorable Monsieur 7 Très bien je mets aux voix cet amendement qui a reçu un double avis favorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté le 141 monsieur le président, Laurent. Oui merci madame la présidente. Bon, il s'agit d'un amendement qui est évidemment un désaccord. Sur une question très importante qui concerne. Le lancement de la construction d'un d'un nouveau porte-. Avions de nouvelle génération. nous mettons en cause ce programme avec cet amendement. Nous savons tous que c'est un. Un programme extrêmement coûteux, donc 10 milliards au total au moins cinq dans cette LPM. Nous le considérons ce choix. Inadaptés opérationnellement face aux nouvelles aux nouvelles menaces. C'est également un outil qui correspond à une conseille une conception de projection de puissance dans les mers lointaines qui n'est pas. Notre modèle. Enfin il a été avancé l'argument selon lequel. Poursuivre ce programme était nécessaire pour assurer la pérennité. De la maîtrise de la filière. Nucléaire Nucléaire en particulier militaires en particulier celle des chaudières nucléaires. Or nous produisons régulièrement. Des nouvelles chaudières nucléaires. Pour les sous-marins. Lanceurs d'engins sans avoir. Besoin de lancer ce ce programme. Donc évidemment, je sais que c'est un désaccord mais je tenais à la à l'ex-. et par cohérence comme ça j'aurais défendu le 142. Évidemment, nous proposons de supprimer l'alinéa qui a été rajouté. Dans le débat à l'Assemblée nationale. Pour lancer des études pour un 2ème porte-avions évidemment par cohérence si nous ne sommes pas pour le premier, nous ne sommes pas pour étudier le lancement du 2ème.

Monsieur Gontard pour l'identique. Ce président Gontard. Vous avez un identique au 142 de monsieur Laurent. Merci madame le président tout à fait. Non ben pour aller dans le sens de ce cas a, de ce qu'a dit Pierre Pierre Laurent. C'est vrai que nous si par contre on est. Pour le renouvellement du porte-avions Charles-de-Gaulle qui arrive en fin de vie et qui semble incontournable. C'est vrai qu'on ne comprend pas tout à fait, on ne comprend même pas du tout cet alinéa qui a été rajouté effectivement à l'Assemblée nationale. Pour adopter une étude de faisabilité pour un autre porte-avions et donc voilà, on est pour la suppression de cet alinéa. Je pense que c'est à la fois absolument pas une priorité qui a d'autres priorités, d'ailleurs dans le domaine maritime. Et d'un contrôle maritime mais certainement pas celle-là, et donc on demande la suppression. La présidente bien évidemment la commission émet un avis très défavorable à cet amendement, le porte-avions futur comme l'actuel le porte-avions Charles-de-Gaulle constituera un atout stratégique et diplomatique majeur pour la France. C'est un outil qui. Pliera des fonctions essentielles, projection de puissance maîtrise des espaces aéro-maritime, mise en oeuvre de la dissuasion nucléaire autonomie d'appréciation des situations. Avec la dissuasion nucléaire. La détention d'un porte-avions et l'un des attributs qui permet à la France de tenir son rang de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies. C'est aussi un atout pour la défense européenne. Il renforce le poids de la France dans le temps et enfin il était un fédérateur de coopération internationale. C'est pour ça. C'est pourquoi le financement du porte-. Avions de nouvelle génération est un point très positif de la LPM et nous émettons un avis défavorable à cet amendement si vous le voulez bien je vais commenter les deux amendements suivants qui visent à supprimer du rapport annexé la demande le lancement d'études de coût pour un second porte-avions de nouvelle génération. La commission est défavorable à ces amendements, c'est quand même intéressant que le Parlement puisse avoir connaissance du coût global que représenterait l'acquisition d'un second porte-avions avis défavorable.

de l'Assemblée nationale. Donc je pense que c'est à vous évidemment de le trouver le raisonnement de vos collègues parlementaires à l'Assemblée nationale était le suivant, c'est plus on va avancer dans le programme du porte-. Avions de nouvelle génération, plus on objectif des coûts qui sont réels et donc c'était pour éclairer la nation disant l'éternel débat du deuxième je veux dire mais au fond, qu'est-ce que ça coûterait vraiment en économie d'échelle en avoir un 2ème et il était entendu qu'il n'est pas question d'en avoir un deuxième donc c'était quelque chose qui tient à la transparence de la structure des coûts. le président rapporteur avec ses collègues députés, voir ce qu'il est bon maître dans la loi, mais je trouve que ça avait du sens qu'il a parfois beaucoup de fantasmes présent comme on a raison de le dire sur les structures de coûts. Du porte-avions et au moins en donnant. Le prix du deuxième et d'ailleurs un certain nombre de vos collègues. Écologistes à l'Assemblée il y était favorable en disant au moins on aura le chiffre aussi non pas favorable au porte-avions ça il n'était pas mais favorable à avoir le bon chiffre pour mieux débattre d'ailleurs donc ça je laisse voir moi pour être transparent demande de retrait sur ces ces amendements. Sur le le le fait de documenter un chiffre parce que d'un côté, on ne peut pas avoir beaucoup beaucoup de demandes au gouvernement comme quoi il faut faire plus de transparence. Éclairer le Parlement sur les grands choix et au moment où précisément les parlementaires à l'Assemblée demande au gouvernement de produire des structures de coûts qu'on aurait jamais donné nous demander de. Si je peux me permettre donc demande de retrait mais ensuite il y a la question du porte-avions en tant que telle. Je pense que le président Laurent va revenir sur les arguments du président Cambon j'aimerais donc tenter d'autres arguments plus militaire. Sur le le l'outil porte-avions en tant que telle. Bon déjà le porte-avions n'existe pas son groupe aéronaval. Donc en fait quand on parle du porte-, avions, je pense qu'il faut le remettre dans son contexte global, c'est le groupe aéronaval. Il repose quand même au-delà même de la faim nu sur les les forces nucléaires sur. Autres font d'ailleurs nous sommes la dernière puissance à avoir une famille donc je j'isole la famille de mon propos, monsieur le président, Laurent. On voit bien que jadis la mer était un espace de conflictualité qui permettait tout simplement de toucher la terre je débarque. Depuis la mer vers la terre je bombarde la Terre depuis la mer pour faire très vite. La mer devient en tant que telle, un espace de conflictualité liberté d'accès. Des routes maritimes et compris civiles c'est vrai sur l'export évidemment par exemple de nos matières premières agricoles. C'est vrai de l'importation par exemple d'hydrocarbures, c'est Suez c'est Babel modèle c'est Ormuz. C'est un enjeu au fond de faire respecter le droit maritime ce droit maritime, là je parle même pas du volet outre-mer dans nos zones économiques exclusives, pas vraiment des grandes routes maritimes. Et on revient à l'amendement de la ministre-Carlotti, sur la Méditerranée. On ne peut pas ne pas voir que la sécurité de l'espace méditerranéen de vieux de plus en plus tendue c'est vrai sous la mer mer j'ai revient pas là maintenant garder. Câble sous-marin protection des oléoducs tout ça tout ça il y a aussi évidemment. Tout l'enjeu de protection du ciel qui est au-dessus de la mer. mer. Avec désormais la sécurité maritime va passer nécessairement par un appui aérien beaucoup plus durci. Donc ça c'est, c'est un argument qui n'est pas. Moi je suis. Je suis aussi prudent d'ailleurs sur le nombre de tonnage de diplomatie et la mer, tous ces arguments-là à mon avis sont son retour Naples sur le terrain purement tactique opérationnel. C'est pas vrai de dire qu'une frégate. Ou des Corvette peut faire le même travail de protection du ciel qu'un porte-hélicoptères par exemple. Et qu'un porte-avions d'un porte-hélicoptères. Ce n'est pas vrai. Le porte-avions des missions qui lui sont propres et qui par la chasse permet justement d'assurer et d'assumer des polices du ciel. Donc ça je pense que c'est un point clé. Si je suis cohérent et un peu provocant, c'est aussi une des gageure de notre autonomie stratégique, y compris dans l'OTAN. Vous avez a le groupe aéronaval américain Bush qui en permanence en mairie en 1000 en mer Méditerranée. Le jour où on a plus de groupe aéronaval Dieu ne plaise. Ben il est clair que vous abandonnez une partie du du segments tactique militaire. Aux Américains pour le faire en Méditerranée. Le faire nous-mêmes c'est aussi notre capacité à pouvoir interagir dans cet espace. Donc je pense qu'il y a plein d'arguments. Qui ne vous convaincre. On peut être pas parce que la position de votre groupe est historique qui est construite et permanente sur le sujet. Mais au-delà des arguments purement géopolitique ou symbolique. Il y a quand même des réalités dans le combat ou des réalités sécuritaire qui pour le coup mérite d'être souligné et qui justifie le porte-avions pourquoi important nouvelle génération et je mettais après mais je pense que ce thème est un des gros thèmes de clivage entre les formations politiques ici comme à l'Assemblée nationale. Donc ça vaut le coup d'éclairer le Parlement avec les Américains, nous sommes les derniers à le faire à propulsion nucléaire. Et pour cause, il nous faut aussi sanctuariser ce savoir-faire et que le savoir-, faire de la propulsion nucléaire que nous retrouvons sur les 2 chaudière du porte-avions c'est évidemment le même savoir-faire que vous retrouvez sur la propulsion des sous-marins nucléaires d'attaque et la propulsion des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins non propulsion ne veut pas forcément dire dissuasion confère les sous-marins nucléaires d'attaque et il faut pas se raconter d'histoires entre nous le savoir-faire industriel Framatome TechnicAtome Direction des applications militaires. Ce qui se passe au Creusot par exemple pour donner un exemple très concret. Bah, savoir faire là évidemment si on fait pas le porte-. Avions de nouvelle génération. Avec les chaufferies nucléaires on a évidemment une rupture de charge importante pour ce savoir-faire et donc on a bu notre autonomie stratégique par ailleurs. Monsieur Roger. Oui. Je je vais presque avoir un, un soutien ferveur du. Ministre de la Défense à l'amendement que j'ai proposé, qui a été retenu par la commission et qui est de dire. Nous, nous souhaitons qu'on étudie la faisabilité au moment où il y aura la grande revue technique du Charles de Gaulle. Si on peut le conserver quelques années parce que nous pensons, je pense Méditerranée en particulier s'il n'y a pas la présence française. Ben il y a les Russes les Turcs et les Chinois qui ont, on le dit pas assez construisent des porte-avions. Comme des pochettes surprise donc ils en font tous les jours, presque donc. On est opposé à ces amendements qui sont présentés, mais on est favorable à l'amendement qui sera présenté tout à l'heure par la commission pour étudier la faisabilité de conserver encore quelques années le Charles-de-Gaulle en Méditerranée uniquement.

on peut savoir à peu près et et donc c'est de savoir si vraiment on a l'utilité, là on est bien sur une étude de faisabilité et puis ce que vient de dire mon collègue juste avant me me fait dire aussi que on a un autre amendement pour réfléchir sur le fait de prolonger effectivement le Charles de Gaulle. Je pense qu'à un moment il faut être cohérent. Je pense que ça peut être une réflexion là que je trouve plutôt plutôt favorable en tout cas de réfléchir. Ah au fait de de pouvoir prolonger ce ce Charles de Gaulle et d'avoir là pour le coup, une étude de faisabilité mais refaire encore une étude de faisabilité

Oui sur l'étude sur le deuxième je note quand même que Monsieur le Ministre, vous dites quelque chose d'un peu contradictoire, parce que vous dites, il faut l'accepter parce que c'est une demande du Parlement, mais moi je clos le débat par avance, surtout en, qu'en tant que ministre sur un 2ème porte-avions précisément ce qui demande cette étude c'est pour ouvrir le débat sur un 2ème porte-avions C'est pas l'essentiel pour moi l'essentiel pour moi, c'est d'abord sur. La question du du du porte-avions. Sur le groupe aéronaval. Une remarque. Un bâtiment comme le porte-porte-avions nécessite beaucoup de moyens pour sa propre défense. parce que évidemment opérationnellement, un bâtiment de cette nature-là. A fortiori si vous vous projetez dans des guerres de haute intensité est un bâtiment extrêmement vulnérables, tout le monde le sait. Donc, ça nécessite de mobiliser énormément de moyens pour la propre défense du porte-avions que nous mobilisons pas ailleurs, donc c'est pour moi discutable et quant à l'argument qui consiste à nous dire que c'est un attribut de puissance. Sur Terre, c'est très discutable d'ailleurs dans des conflits de bien moins grande intensité. C'est pas parce que nous avons un porte-avions que nous avons réussi à marquer des points en Afrique avec Barkhane et en mer. Par exemple, nous avons joué un rôle très actif et positif

et puisqu'hier, on a fini le débat sur beaucoup sur la question des choix qu'on avait à faire, nous effectivement nous préférons faire des choix d'équipement renforcée des forces dans toute une série de domaines, plutôt que celui du porte-avions pour, je le rappelle quand même 10 milliards d'euros. Y a-t-il d'autres explications de vote avant que je donne la parole au ministre. le porte-avions de de nouvelle génération. Il ne s'agit pas d'un d'un 3ème porte-avions. Il s'agit effectivement de voir si nous aurons la possibilité de maintenir le Charles de Gaulle, au moment de de l'arrêt technique qui sera réalisé à l'échéance 2027 2028 mais je crois qu'il est important de rappeler que même si ce n'est pas un bâtiment de de puissance. C'est en tout cas un bâtiment qui sert à la fois la crédibilité de la nation, mais aussi à la diplomatie. Donc je crois qu'il est, il est important de, de rappeler que lorsque le Charles-de-Gaulle est positionnés en Méditerranée orientale. Les relations entre les États riverains de la Méditerranée ne sont pas les mêmes que lorsqu'il est dans une autre zone du globe et que l'on peut facilement. Crédibilité et diplomatie. Monsieur le Ministre, je n'y a pas d'autre explications de vote. Merci madame la la présidente. Bon, l'argument sur la diplomatie il s'entend complètement Et justement puisque aux opposants au porte-avions j'aime bien y rajouter quand même l'argument purement opérationnel et militaire. Et en fait on ne peut pas s'en sortir. Monsieur le président Laurent en disant on ne fait pas le porte-avions parce qu'on a d'autres besoin d'outre-mer. Déjà pardon parce que la marine nationale remplit les objectifs qui lui sont assignés, en outre-mer on peut toujours faire plus mais si il y a plus le porte-avions il est certain que l'émission qu'on affecté au porte-avions ne pourra pas les assumer autrement en Méditerranée et ça, je pense aussi qu'il faut qu'on l'assume. On ne peut pas ne pas voir les dîners d'accès. Que nous avons sur certaines routes maritimes notamment liés à l'Iran pour dire les choses assez directement. Et se dire qu'une puissance comme un autre, pas pour des raisons diplomatiques, mais va abandonner un certain nombre de missions opérationnelles. Quand on dit diplomatie c'est pas que du signalement. Un porte-avions un groupe aéronaval c'est comme un gros bloc multiprise dans lequel ça nous permet d'emmener d'autres quand le groupe aéronaval du Charles de Gaulle ce dépôt en Méditerranée. C'est comme ça que vous avez une frégate grecque. Une corvette italienne enfin on fait aussi ce qu'on appelle une forme de nation-cadre maritime dans lequel on est capable d'agréger et pas agrégé pour faire du signalement diplo ma tique mais agrégé pour muscler une capacité entraîner et si je suis honnête avec vous, c'est ce que je ne comprends pas dans la position du groupe communiste contre le porte-avions c'est qu'il est fondamentalement contraire à ce que vous voulez par ailleurs faire en sortant du commandement intégré de l'OTAN. Parce qu'en fait, dès lors qu'on sort du commandement intégré de l'OTAN. Si on suit votre logique. Il est clair qu'il faut qu'on ait des capacités d'entraînement propre. Et il y a pas de doute, enfin je veux dire si on fait pas de multilatéral dont l'intégrer dans le commandement intégré de l'OTAN ou dans le Ben faut bien quand même trouvé le moyen de faire du multilatéral militaire autrement. Donc en fait je, je sais, ça je l'ai dit à vos collègues aussi à l'Assemblée. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est antinomique entre la volonté de sortir du commandement intégré et en même temps de se priver l'outil porte-avions il y a quelque chose qui, qui fonctionne pas bien de. Pour le président Gontard non. s'il y avait un 2ème porte-. Avions de nouvelle génération, il ne serait pas du même coup que le premier et nous ne savons pas donné le coup aujourd'hui. C'est d'ailleurs le le l'argument des promoteurs d'un 2ème porte-avions qui est de dire, mais voyons tout ça n'est pas suffisamment Challenge et il y a des coûts de structure si vous en avez fait hein c'est que le 2ème coûte moins cher parce que vous amortissait le prix des études et cetera et cetera c'est comme ça que vos collègues à l'Assemblée on dit bah si vous n'avez rien à cacher. Dites-nous le montant au moins ont conscience, on verra qu'on ne peut pas se le payer. Trois oui je l'évacue d'autorité. Dans le cas de la programmation militaire que je vous propose pas commencer entretenir une ambiguïté, il y a pas de 2ème porte-avions financés dans cette affaire et de pour la raison que vous avez vous même pointé monsieur le président, Laurent. Un porte-avions n'est rien sans sa garde son son groupe aéronaval et donc s'il devait y avoir un 2ème porte-avions c'est par définition l'augmentation à du concurrence du nombre de sous-marins nucléaires d'attaque des équipages. Des frégates qui vont bien de la guerre des mines évidemment qui va autour, c'est pas le sujet. Donc il ne faut pas caricaturer ce qui a été intégrée par vos collègues parlementaires à l'Assemblée de documenter le prix de quatre et ça me permettra de revenir à l'amendement du groupe socialiste qui arrivera plus tard dans la discussion sur l'avenir du Charles-de-Gaulle, on sera peut-être amenés à si vous en êtes d'accord à adapter l'amendement que vous déposez. Il y a une inconnue qu'il faut qu'on assume collectivement dans la programmation, c'est à la prochaine arrêt technique majeur du Charles-de-Gaulle Carole ont 28. Cet arrêt technique majeur mais comme un arrêt technique sur une des tranches de centrales nucléaires diront des choses des de chaudière et plus encore des 2 cuves et pourront permettre aux autorités du moment de prendre des décisions sur le calendrier de fin du Charles de Gaulle et ça, si vous en êtes d'accord, tout à l'heure là il est écrit dans l'amendement. Je crois que dans les six mois il faut qu'on puisse vous le on ne saura pas le faire dans les six mois parce que c'est l'heure de l'arrêt technique majeur qu'on pourra lire mais je pense que pour le coup on programme bien en disant qu'en 2028 en fonction de ce qui se passera sur l'arrêt technique majeur, le ministre-du moment viendra devant l'Assemblée et le Sénat du moment pour dire ce qui se passera pour le Charles de Gaulle, donc tout à l'heure si vous êtes d'accord monsieur sénateur on prendra l'amendement en le corrigeant quelque peu pour le rendre complètement voilà sur l'ensemble du débat sur le portable. Très bien je vais donc mettre aux voix d'abord le 141 d'avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté. Le 142 220 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés. Nous passons monsieur Folliot à l'amendement 22. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, vous avez toujours dit, c'est une position constante de la France. De veiller à ce que nous puissions assumer un certain nombre de missions et notamment. Le respect du droit international et la liberté de navigation. Il y a une zone très sensible. À travers. Le monde par rapport à cela. C'est plus particulièrement le Detroit de Taïwan.

à envoyer une R 16 sur une autoroute fréquentée par des 38 tonnes flambant 9 américaine et chinois pour symboliser les choses. Au travers de cet amendement. En fait, je vous propose à ce que, à compter de 2030. Toutes les affectations que nous aurons plus particulièrement les nouveaux moyens. En 2 frégates de 1er rang, il puisse y avoir un prépositionnement dans nos outre-mer. Pour 2 raisons. La première c'est pour être conforme à ce que j'ai défendu ce que je défends, c'est passé d'une logique de de moitié, Brest, Toulon, à une logique des quatre car, Brest, Toulon, Saint-Denis. Pour l'océan Indien Papeete ou Nouméa pour le Pacifique, avoir une meilleure prédit prédispositions. Et prépositionnement de nos moyens. De 1er rang au niveau de la Marine nationale le second. Imaginons un moment. Que pour une raison ou pour une autre, nous ayons des relations avec l'Égypte et Panama, qui font que ces deux Canal soit fermé le temps de d'envoyer des moyens de l'Hexagone va poser quand même beaucoup de difficultés. C'est pour cela que un pré-positionnement de moyens de 1er rang au niveau de la marine nationale dans nos Outre-mer et quelque chose d'important et des syndicats. La commission a pris bien évidemment la la mesure et approuve le souci de renforcer les moyens de la marine nationale outre-mer. Néanmoins, il ne nous revient pas de décider maintenant de l'affectation de bâtiments qui seront éventuellement comme après 2030. Donc je ne suis pas personnellement favorable à ce type de priorisation systématique car la marine. A et aura bien besoin de souplesse dans la gestion de ses moyens, notamment en cas de tension croissante dans l'indopacifique Merci madame présentement c'est un amendement d'appel parce qu'effectivement faire de l'affectation dans une programmation pour des bateaux qui n'existe pas encore. Par définition, c'est pas possible. 2ème argument c'est évidemment l'état major des armées de faire des propositions, le cas échéant trois plutôt que d'affectation va surtout falloir compatissent l'émission différemment et vous qui connaissez bien cette affaire, vous voyez ce qu'on en train de faire avec Pégase est un véritable changement opérationnel l'avantage nous des nouvelles technologies, des nouvelles générations de matériel, y compris pour les avions, on le voit bien avec Pitch Black en en Nouvelle Calédonie. Bah vous nous autorisez aussi à avoir des projections temporaire mais récurrentes qui vont être quand même très précieux sur un certain nombre de sujets après si on raisonne mais les marins vous le diront mieux que moi affecté une frégate que quand même un, un objet particulièrement lourd en permanence à un territoire d'outre-mer aujourd'hui ne couvrirait aucune menace réelle enfin sauf à à vouloir être aimable mais heureusement aucun territoire d'outre-mer n'est confrontée à un risque militaire qui nous mettrait à devoir mettre une frégate en première ligne et puis si j'en Léa si vraiment on avait un risque militaire de cette nature, on serait amené à avoir un niveau de réactions qui de toute façon ce serait bien nous de là. Si vous voulez, ce que je veux dire qu'une seule frégates donc demande de retrait sachant que dans les amendements qui viendront, on y reviendra mais il y a peut-être des choses qu'on peut qu'on peut retenir sur le le volet réflexion et innovation. Merci. Monsieur Folliot, vous voulez. Sur votre amendement. Oui. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Bon je vais retirer cet, cet, cet amendement mais je voudrais simplement, Monsieur le Ministre vous dire une chose. comme vous dites par rapport aux enjeux relatifs au prépositionnement. Et au regard des menaces ce qu'il peut y avoir par rapport à nos outre-mer il sait pas du tout la même chose en fait, ce que je propose et ce que je suggère au travers de cet amendement. C'est le fait d'avoir un prépositionnement dans le cadre d'une stratégie indopacifique qui ferait que c'est pas la même chose quand vous avez des moyens qui sont prépositionnés dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique que quand vous envoyez même pour des missions qui sont organisés structurés préparé de de de de longue date. Vous avez parlé de Pégase et de l'équivalent qui pourrait être fait au niveau de la marine nationale. C'est pas du tout la même signification politique par rapport à un autre environnement géostratégique. Que d'avoir des moyens prépositionnés que d'envoyer des moyennes de l'Hexagone. de de de de cet amendement et de ce que j'essaye de défendre visiblement avec pas assez de conviction mais en tout état de cause qui me paraît important et essentiel par rapport à ces enjeux.

et à la préservation donc. De de notre souveraineté, notamment au niveau des Outre-mer mer. Nous savons que le nombre de patrouilleurs et est largement. et que par rapport à cela. En fait. Ce qui est ce qui est fait tout juste suffisante pour répondre aux besoins et donc. Cet amendement vise à ce que une étude complémentaire sur le nombre de patrouilleurs nécessaires à la protection et à la surveillance effective de notre domaine maritime ultramarins se ramener les éventuelles unités qui pourraient être commandés devront suivre un schéma de répartition fixant une priorité à l'affectation dans l'Outre-mer des nouvelles capacités. Je crois que cette. Un point qui est un point est essentiel juste rappeler. 97,5% dans notre zone économique exclusive est lié aux Outre-mer. Hampton 95% des moyennes de notre Marine nationale sont basés dans l'Hexagone. Il y a tout juste un problème et que par rapport à cela il faut que nous puissions avancer et un autre point, Monsieur le Ministre. Alors tout le monde ne serait déçu si je n'en pas mais c'est par rapport à l'île de la passion, Clipperton et et on regarde du fait que le contrat opérationnel, tel qu'il est fixé aujourd'hui. Dit que tous les trois ans. La marine nationale doit aller dans la zone économique de l'île de la passion qui perd, qui avait 436.000 km2 plus importante que celle de l'Hexagone Corse comprise qui fait 345.000 km2. Comment est-on crédible et comment peut-on raisonnablement assurer la souveraineté en allant une fois tous les 3 ans sur une partie du territoire national, ça interpelle et que donc le fait d'avoir d'autres moyens et des moyens plus importants prépositionnés donc. Dans. Le Pacifique et en Polynésie nous permettra d'assurer une souveraineté un petit peu plus effective en attendant. De scientifique. Alors l'île de la passion Clipperton.

Passionnant mais c'est vrai qu'il faut s'en occuper et je l'ai dit en commission. Donc tout ce qui concerne tout ce qui va dans le sens d'un renforcement de nos moyens. Est évidemment favorable est vu favorablement Léon néanmoins cet amendement pose quelques problèmes notamment. La demande d'une étude complémentaire sur le nombre de patrouilleurs nécessaires puis après l'amendement semble préjuger de la conclusion de l'étude qui a été demandé en priorisant les outre-mer dans l'affectation des nouveaux patrouilleurs éventuels. Je crois que le message est bien entendu je propose à notre collègue de de retirer cet amendement, faute de quoi il aurait un avis défavorable de la commission. Oui. J'ai compris, il faut que je fasse vite. Mais non mais j'ai un est illimité mais madame la ministre-présidente. Je comprends que vous soyez vigilantes autant de parole y compris du ministre, même s'il est illimité. Je suis donc télégraphique et rapide j'ai j'ai du mal avec les arguments sur le tonnage à la mer parce que ça peut nous faire mal raisonner à l'avenir. Confère spatiale drone dont on a besoin pour les outre-mer. Or le poids d'un drone par rapport au point d'un bateau sur la surveillance d'une économie je cuisine ou le point. Un satellite par rapport au point d'un bateau, j'en fais exprès en disant ça mais comme vous l'avez injectée mais ben si mais quand même. attendez dans toute la construction va en plus que je je le regarde un de mes prédécesseurs désormais. Savoir Gérard Longuet qui nous a rejoint. Il est clair que la la le la volonté de mettre plus de tonnage d'acier à la mer n'est pas le seul gage de sécurité dans l'émission de la marine nationale de demain. Voilà et d'ailleurs le chef de la Maison de la marine, vous l'a dit, c'est pour ça qu'on a une copie particulièrement allante sur les moyens aériens de la marine nationale parce que pour le coup sur les mesures de surveillance en outre-mer mer notamment. C'est aussi par les airs que les choses se font. Première remarque. 2ème remarque dans la copie vous avez la première Corvette hauturière dans la période qui n'étaient pas prévus dans la LPM précédente parce que justement ça répond aux besoins que vous avez identifié, il est clair que sur la LPM 2032 1035. À mon avis il faudra poursuivre le moment venu cet effort, la 3ème chose. un, un souhait de l'Assemblée nationale que de rentrer les études pour essayer de faire justement émergé ce segments bien connu jadis mais sur un segment en un peu plus dur parce que si on est sur une mer un peu plus agitée ou un peu plus, un peu plus en haute mer. Il faut quand même évidemment avoir déjà des équipements qui ont des tonnages suffisant et donc là aussi pour le coup ça été satisfait par ce qui a été injecté par l'Assemblée nationale. On demande de retrait. Monsieur Folliot vous retirer. Vous maintenez. D'accord donc je mettre voix cet amendement 23 qui a reçu un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 28 c'est vous monsieur

Qui est la seule capacité qu'un autre pays à pouvoir aller dans les grandes font puisque la France fait partie. Des rares nations qui maîtrise c'était technologie et cette capacité à pouvoir aller dans les grandes font. À 6000 mètres qui est qui est qui et qui me semble important de sauvegarder. D'autant plus, on va pas revenir sur l'actualité très récente au travers du drame qui s'est passé, que tout le monde un mémoire mais au-delà de cela. La décision. De l'Ifremer a été de dire nous allons arrêter le Nautile à partir de 2028 pour un million d'euros par an. D'économies de budget c'est-à-dire que la France va sortir de la capacité des nations à pouvoir. Aller dans les grands fonds pour faire une économie d'un million d'euros par an. Et la question qu'on peut se poser, c'est le but de cet amendement. C'est un homme de dire après tout ces enjeux. Relatives aux grandes sont des enjeux du au civil. Regarde la recherche et cetera mais aussi militaire. Nous le voyons et les uns et les autres par rapport à une capacité que nous pourrions avoir. En observation et que les drônes sous-marins ne pourront pas tout faire. Et de la même façon et donc pour conserver cette capacité à pouvoir. Aller dans les grands fonds pour faire de telle sorte que celle-ci puisse être complémentaires donc et dual, civil et et militaire. Il me paraît important d'inscrire donc dans cette loi de programmation militaire. Le fait que. La France. Essayera de maintenir sa capacité donc avec un partenariat qui sera un partenariat. Civil, militaire public-privé pour maintenir donc le Nautile et son successeur. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le président. Bon. À la Commission va donner un avis favorable à cet amendement parce qu'il s'agit de mutualiser le sous-marin habité le Nautile de l'Ifremer, avec les armées. La stratégie de de maîtrise des fonds marins du ministère des Armées se concentre sur l'acquisition de véhicules autonomes non habité capable de descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur et dans l'attente du développement de capacité souveraine des drone norvégiens sont actuellement testés par la marine nationale. Or la France effectivement dispose de compétences historique dans ce domaine des grands fonds marins notamment grâce à l'Ifremer et à la flotte océanographique française. Ce qui a permis de déployer le Victor 6000 récemment déployés pour tenter de porter secours au submersible porté dramatiquement disparu près du Titanic. Alors l'Ifremer dispose également du Nautile sous-marin habité capable de plonger à 6000 mètres, ce, ce Nautil ce sous-marin habité a permis du reste de de très nombreuses découvertes scientifiques. Or, la Marine nationale ne dispose pas en prof d'une telle capacité et comme ce, note-t-il, constitue une ressource rare, on ne peut que encourager sa mutualisation civilo-militaire, un avis favorable. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, non. Avis favorable avec une demande de rectification. C'est le changer d'endroit. Si vous en êtes d'accord dans le rapport annexé. Il y a un paragraphe dédié au fonds sous-marins et à l'innovation. Là ça va se mettre en note de bas de page sur le tableau capacitaire donc. On vient de regarder si vous acceptez de le rectifier pour le mettre à. Dans le paragraphe fonctionnement la lignée 33 après la sixième phrase mais le même texte. Votre amendement. À l'identique mais au bon endroit.

Nous allons voter contre cet amendement. Qui est significatif. Ah du risque que je vois à devenir concernant la militarisation. De nos politiques dans les fonds sous-marins et dans l'espace, parce qu'on gros à l'argumentation consiste à dire que. Nous laissons disparaître des capacités civiles. Dans l'indifférence générale. On va arrêter le Nautile. Et puis maintenant on va on va le mettre dans une situation d'utilisation duale, civile, militaire et donc là on peut mettre de l'argent le sauver mais ça a une conséquence parce que quand c'est l'Ifremer qui travaille l'Ifremer. Elle travaille comme nous le faisons dans l'espace civil en coopération ouverte. Comme c'est la règle de la coopération scientifique internationale. Si nous assignant des fonctions militaires à ce bâtiment alors ses fonctions seront restreintes en matière de coopération internationale. Par définition, puisqu'en partie couverte par. Les, les règles de la non-coopération militaire sauf avec des alliés mais pas forcément avec d'autres nations et etc donc nous passons d'une situation, nous avons un bâtiment qui fait de la coopération internationale ouverte. Un bâtiment qui lui va le faire de manière. Considérablement restreinte et c'est à ça que risque de conduire et la militarisation de l'espace et la militarisation. Dans les les fonds sous-marins c'est extrêmement inquiétant et je trouve que cet exemple d'une autre, il est particulièrement significatif de ce risque. Donc moi je serais. Pour effectivement qu'on garde le le Nautile à faire son travail mais mettons 1 million de plus dans la recherche civile pour pouvoir le faire mais pas au militarisation pas aux militaires à raison. Sa fonction, avec les conséquences que cela aura. En matière de fermeture de coopération scientifique internationale. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, je dirais qu'a contrario de l'argumentation développée à l'instant par le président Laurent je dirais qu'au contraire il faut que l'on développe les synergies notamment de recherche entre le civil et le militaire. Il est bien évident que. Nous avons des intérêts communs pour faire progresser l'activité industrielle dans notre pays, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays, je pense à la Norvège que la mission dédiée aux fonds marins avaient pu. Rencontrer des interlocuteurs Norvège se rendent compte comme. La synergie des actions de recherche. Liées à des secteurs qui demande des évolutions technologiques extrêmement performante. Pouvait amener au développement d'outils intéressants à la fois le civils et militaires donc. Je crois qu'. Il faut au contraire que nous puissions encourager ce genre de démarche et tenir compte des besoins d'Ifremer pour le renouvellement du Nautile qui est un outil aussi particulièrement important. On le voit bien à l'aune de ce que nous avons. Connues sur les accidents marin très récemment je me l'océan. Bien je vais donc mettre aux voix monsieur

Un outil éventuellement de renseignements pour voir pour. Regarder un certain nombre de choses par rapport à des câbles ou autre, mais en tout état de cause n'a pas de capacité d'une manière ou d'une autre à pouvoir mener des actions qui soient des actions agressives létale ou quoi que ce soit à l'égard de qui que ce soit, ça restera un outil d'observation. Merci bien. Comme il n'y a plus d'explications de vote, je vais mettre aux voix cet amendement 28. Réécrit par sur proposition du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Nous avons maintenant le 167 monsieur Folliot. Oui merci. Madame la présidente. Cet amendement vise à essayer de faire de telle sorte toujours par rapport au aux outre-mer. Hein. Donner une forme de priorité par rapport à l'équipement de drone. Donc au niveau de l'ensemble des bâtiments parce que tout un chacun a compris que, un, un, un bâtiment a une capacité de surveillance de visu ou de radars qui est ce qu'elle est mais un drone, notamment pour ceux qui n'ont pas la capacité, la possibilité d'embarquer des hélicoptères donnera une capacité d'allonge je pourrai aller voir

association d'affectation donc des des drone au fur et à mesure que ceux-ci seront mises en service. Donc dans les bâtiments de la Marine nationale, et plus particulièrement. Donc ce qui exerce ses missions de souveraineté outre-mer je crois que c'est un enjeu important par rapport à la lutte contre les trafics par rapport à la problématique. De la préservation des ressources halieutiques. Par rapport à tous les enjeux de défense de l'environnement en fait toutes les missions. Qui sont celles de surveillance faites donc par. Nos différents bâtiments patrouilleur ou frégates de surveillance. Ultramarines. Alors la Commission regarder de près cet amendement et. Le, je rappelle que le rapport annexé programme dit système dit système. Désert, ces systèmes de drônes aériens pour la marine. En 2030 l'atteinte de l'objectif de 15 est reporté à 2035 et ce chiffre correspond au nombre de frégates de 1er rang de. Par ailleurs le dame peut être utilisé sur d'autres types de bâtiments. Donc il faudrait probablement une trentaine de systèmes pour atteindre l'objectif de cet amendement, ce qui nous paraît difficilement réalisable. Et par ailleurs il nous apparaît aussi beaucoup trop d'prescriptif quant à l'usage par la marine de ses moyens. Donc je propose. À Philippe Folliot, soit de retirer cet amendement. L'appel est entendu, sinon l'avis est défavorable. Monsieur le Ministre mais mais oui mais présidente. Monsieur Folliot, vous maintenez. merci. Monsieur Bono pour le 44. En exergue, comme il a été dit dans le rapport d'information sur, sur la guerre des drone et se préparer à celle-ci comme enjeu stratégique. L'utilisation massive de de de ses 20 Drôme comme on a pu le voir dans les différents conflits et malheureusement le conflit actuel donc. Il s'agit au regard de ce. De cet amendement n'ont pas de demander une dépense supplémentaire de rester dans l'enveloppe mais. S'agissant de de ces drone de prévoir une dotation suffisante en drone que l'on appellerait ça crée fiable. Armés ou non armés afin de s'adapter aux nouveaux modes opératoires qui qui se déploie aujourd'hui. Merci, qui a de l'avis de la commission. Un président de cet amendement est en fait de satisfait par l'adoption de l'amendement 124 de notre collègue Cédric Perrin qui est beaucoup plus ambitieux puisqu'il programme au moins acquisition de 1800 munitions de ce type. Donc je propose notre collègue de retirer cet amendement, faute de quoi l'avis serait défavorable. Même ma vie madame le président. Merci Monsieur le Ministre, Monsieur Bono. Il n'y retiré. Le passant 21 monsieur Folliot s'est de nouveau à vous. Je vous rassure, madame la présidente. Et je je. Ça c'est cet amendement. Pour être en cohérence avec ce que nous défendons que se défendre et que nous défendons au groupe Union centriste. de de de la volonté de prépositionnement. Donc de nos, de nos forces. Et et au regard aussi du fait de maintenir comme nous l'avons dit dans le cadre de la discussion générale, une capacité de projection mais que c'est pas capacité de projection sont aujourd'hui toutes basées dans l'Hexagone et donc en fait il s'agit au travers de cet amendement de dire. Des priorités. D'affectation donc. Des futurs A 400 M que l'aspect d'équilibre avec nos outre-mer et notamment toujours pour en revenir à nos éléments de stratégie par rapport à l'Indopacifique. Mais n'oublions pas aussi. Les enjeux relatives aux Antilles Guyane où les seuls moyens que nous avons aujourd'hui au travers de Casa puisque les Transal ne ne ne sont plus. Donc en service s'avère souvent assez limité et donc ça c'est le 1er point par rapport à des enjeux territoriaux locaux mais aussi, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure Monsieur le Ministre, par rapport à la notion d'image. Au niveau de la France de rayonnement pour notre pays au travers donc de la capacité, par le biais de ses avions et et comme vous l'avez fort justement dit souligné dans le cadre de l'opération Pégase mais M. va aller à de Nouvelle Calédonie de la Nouvelle Calédonie. Je crois qu'il est prévu un certain nombre de missions aux Fidji et et dans les pays environnants et bien finalement. Une posture qui est utile mais qui va être temporaire, hé bien nous proposerons qu'elle devienne permanente par le biais du vote de cet amendement. Monsieur le Président quand bon. La Commission va rendre un avis favorable sur cet amendement car. Certes le projet de LPM fixe un objectif d'au moins 35 aéronefs au lieu des 50 qui était prévu dans le cadre de la LPM actuelle. Alors bien sûr, une augmentation plus substantielle de la flotte pourra être pourra être envisagée non seulement bien sûr pour préserver le programme export mais surtout pour répondre à un besoin de projection notamment vers et à partir l'outre-mer Philippe il faut lui a souligné. Les les exploits. Que que a pu. Réaliser notamment dans les opérations de rapatriement à partir de la Polynésie française. Sont larges. Son large rayon d'action, le rend particulièrement adaptée au contexte de l'indopacifique. Alors bien sûr il faudra que cet amendement soit poursuivi par une étude et par ailleurs, il faudra une adaptation des infrastructures pour faciliter ce genre d'opération. Avis favorable. Monsieur le Ministre. Bien la présidente. Malheureusement, j'ai envie envoyé il y a pas besoin d'étude, c'est une affaire désormais d'enveloppe. Donc, je ne commence pas le débat, nocturne donc défavorable. Cet amendement qui a reçu un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté le 283 monsieur le ministre. Oui mais la. Il est défendu et je mettrai tout de suite un avis de sagesse sur le sous-amendement monsieur Perrin. Je pense que ça éclaire le Sénat dans le sens des débats, des questions qui m'avait été posée en commission.

N'ayant pas eu le bonheur de participer à la. Travaux de la commission. Je voulais savoir quel était le point de vue du ministre sur le maître d'ouvrage de ce. Éléments de combat lourds terrestre. Parce que nous sommes, par l'intermédiaire de cas une déesse associée aux Allemands de cross ma faille qui ont eux-mêmes leurs propres projets étant les héritiers je crois. De la. Lignée. Léopard dans quel, pouvez-vous nous éclairer sur ce point. Il va le faire. Merci. Madame la présidente, monsieur Ministre. Pour de fait la l'amendement évidemment c'est sur la rénovation du Leclerc sujet entendu éclairé, j'y reviens pas. Votre question c'est le le jour d'après. Du Leclerc je pourrais éclairer le Sénat et repartir du début. Exactement mais pour parce qu'en fait c'est comme pour le SCAF, on finit par penser que. On va du Rafale au au Skaf et on finit par oublier qu'il a un standard quatre et un standard

dans lequel l'Allemagne et chef de file comme nous sommes, chef de file sur le SCAF avec des discussions actuellement franche avec. Le partenaire allemand, quand je dis franche le partenaire, c'est le ministère de la Défense entre États. Sur déjà le cahier des charges de ce qu'on attend de ce char. Quand je dis de ce qu'on attend c'est ce qu'on attend militairement puisque le 2040 offrent quand même. Des réflexions qui sont assez larges et ce qu'il est habité, ce qui n'est pas habitée, s'il est habité ce qu'il est encore habité de 4 cavaliers comme aujourd'hui, ou au contraire opérer de manière différente, est-ce qu'au contraire on est sur un, un, un modèle qui est un peu plus hybride qu'est la part de guerre électronique et de drone ou drone ou de Claude qui est autour du donc déjà il y a un 2ème. Discussion qui est actuellement en cours, c'est entre les deux chefs d'état major des 2 armées de terre, les deux pays pour s'assurer déjà du cahier des charges. Du client final, à savoir les deux les deux ministères. Je le précise parce que c'est ce que nous avons exigé pour le SCAF et donc nous l'exigeons aussi évidemment pour le MGCS 3ème les choses. Le montage industriel et nous on arrive à votre question précise. Il est clair que qu'NDS. Doit être au coeur du du programme pour nous. Moi je défends le savoir-faire de cas une déesse en la matière, ici ou là dans la presse on pourrait lire que Rheinmetall serait peut être meilleur que que NDS sur certaines fonctions, notamment le feu et je pense qu'il suffit de regarder le succès du canon Caesar actuellement pour voir que. Les savoir-faire français en la matière sont absolument remarquables. Je précise aussi que si cas NDS évolue dans le format que vous connaissez dans sa filiale ou en tout cas dans sa branche française dans sa branche allemande, c'était aussi pour faire évidemment ce ce projet et donc pour nous il est très clair que le programme doit se faire avec NDS. Voilà en quelques mots, si vous avez d'autres éléments, évidemment, je suis à votre disposition. Je vais donc mettre aux voix cet amendement du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Madame Conway Mouret pour le 88. l'Intelligence artificielle ou IA est une technologie de rupture dans laquelle nous devons investir dès maintenant pour ne pas être distancié surtout c'est un sujet dont nous n'avons pas beaucoup parlé dans ce texte, et dans son examen alors qu'elle s'impose à nous, dans tous les domaines. Pour ce qui relève de la défense, je pense qu'un, un débat sur l'éthique de son utilisation s'impose. Et puis européens ont déjà pris du retard alors que les trois quarts des brevets en matière d'IA déposé entre 2010 et 2022 sont américains, seuls 2,4% sont français. L'Intelligence artificielle représente pourtant un véritable enjeu de souveraineté, d'une part le manque de financement pour les entreprises européennes à s'installer de l'autre côté de l'Atlantique en 2021 la Banque européenne d'investissement avait estimé à 10 milliards d'euros le déficit annuel d'investissement de l'Union européenne Dans LIA à de comparaison la Chine ambitionne de devenir le leader mondial et investit 1,6 milliards d'euros par an dans l'IA contre 100 millions d'euros par an pour la France. D'autre part l'hypothèse selon laquelle un locataire de la Maison Blanche interdirait l'utilisation de certains outils américain n'est pas non plus à exclure. Elle représente également un enjeu stratégique opérationnel voire tactique en triant et classifiant un énorme volume de données il y a permet à nos armées d'anticiper et leur confère une supériorité informationnel in fine, elle permet d'améliorer les conditions d'engagement de nos forces pour toutes ces raisons, l'Intelligence artificielle devait très devrait être considéré comme un programme à effet majeur. Mes chers collègues, l'amendement qui vous est proposé, a pour objectif de marquer la prise de conscience par le Parlement des enjeux, que représente la généralisation de de l'IA au service de la Défense ainsi que des investissements nécessaires pour maintenir notre rang face à la concurrence internationale. Je vous remercie. et donc ça c'est tout à fait intéressant. Avis favorable. Monsieur le Ministre. Oui merci beaucoup. Mais alors c'est pas le rapport annexé qui ouvrent la ligne budgétaire, de toute façon elle est déjà elle est déjà prévu, néanmoins tout ce qui est dit en matière de doctrine sur l'IA correspond à ce que nous souhaitons faire donc avis favorable Madame la Ministre. Très bien, je vais mettre aux voix cet amendement 88 qui a reçu un doublé favorable qui est pour. Qui compte qui s'abstient adopté de de 73 du gouvernement. Oui il est défendu et d'un mot pour moi, c'est l'exemple concret où il ne faut pas introduire trop de rigidité justement dans la programmation. La chronique des crédits en matière d'innovation. Elle est dans la copie, elle est beaucoup délégué à la DGA et notamment la idée et donc par définition elle est dans la programmation. La chronique annuelle à mon avis n'a que n'a que peu d'intérêt. D'où l'amendement du gouvernement qui vous est proposé. Monsieur le Président quand bon quel est votre avis. Ça j'ai sur cet moment sagesse. Je vais donc mettre aux voix cet amendement de monsieur le Ministre. Et dans le retour de la sagesse de la commission. Il va sans dire que dans la mise à jour. Et la programmation annuelle lorsqu'on est avant la loi de finances. Si le Sénat a besoin d'informations sur les crédits qui sont proposées en matière d'innovation, le gouvernement il transmettra c'est l'engagement que je voulais donner au. Merci je mets aux voix cet amendement du gouvernement qui a reçu un avis de sagesse de la commission qui est pour, des contres qui s'abstient adopté monsieur Perrin ne 162.

Il est nécessaire aujourd'hui de gagner en agilité en rapidité. L'acquisition d'où l'idée que nous avons intégré. Dans la loi de programmation militaire de concevoir un système de drone de confiance ce système de drone de confiance il aurait pour objectif notamment. De faire un petit peu une méthode d'acquisition à l'identique à celle que l'UGAP met en oeuvre pour les collectivités notamment pour pouvoir être beaucoup plus rapide et beaucoup plus Agile et pouvoir surtout obtenir des drone qui soient sécurisés et validé. En amont, peut-être par l'Anssi enfin tout ça reste à déterminer la manière dont on dont se doivent être faits, d'autres, restait à déterminer mais ce qui me paraît important c'est que. Les autres services de l'État je parle là pour le. Monsieur le Ministre et je pense que c'est un point important, les autres services de l'État puisse bénéficier de l'expérience et de l'expertise désarmés. Parce qu'il y a quelques points qui me paraissent moi particulièrement inquiétant et j'ai juste je vais vous donnez un élément qui vient de la préfecture de police de Paris, c'est le service de sécurité intérieure. Mais je pense que un système de drone de confiance pourrait aussi bénéficier au service de sécurité intérieure qui explique qu'ils utilisent des drônes de marque que je ne citerai pas chinoise leader sur le marché dès au au plan technique, qui sont des drone qui ne sont pas modifiées. Le risque d'espionnage et réduit car les engins doivent être connecté à Internet pour transmettre des informations et nous sommes en mesure de contrôler cette connexion. De plus, les images captées par les drone ont un intérêt local très limitée, donc pas de problème, je pense que ça résume en quelques mots. Je pense en tout cas l'incompréhension de la problématique du cyber de de la de la sécurisation de nos drônes. Donc, ce système a pour objectif d'être Agile et de gagner en rapidité et surtout en efficacité en matière de sécurisation et donc le présent amendement demande à ce que ce dispositif soit finalisé d'ici à la fin de l'année 2024. Merci. Monsieur le Président quand bon. Qu'en pensez-vous. Favorable, Favorable, Monsieur le Ministre, sagesse, sagesse jamais aux voix cet amendement avis favorable du gouverneur de la commission et sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté cet amendement faisant l'objet d'une édition commune. Avec un amendement 274 du gouvernement. Et là il y aura trois sous-amendements. Alors l'amendement est défendu et ce sera un avis favorable pour l'ensemble des sous-amendements qui viendront, je me permet de faire une fois comme ça ça va. Et dès la présentation intellectuellement des choses. OK alors. On va quand même demander à monsieur Perrain défendent son sous-amendements le 307. Très très rapidement. Cette histoire a commencé à être ancienne puisqu'au moment du de la décision en septembre 2017 de la précédente Ministre des Armées d'armer les drônes Reaper. Nous avions oublié peut être de demander l'armement des des pas trop leur aujourd'hui c'est quelque chose qui est dans les tuyaux mais qui met un peu de temps donc on demande tout simplement ce que ce soit accéléré parce qu'évidemment c'est un sujet particulièrement important et donc l'armement des 28 drone tactiques pas trop leur inscrit à la loi de programmation militaire est un sujet. Que nous attendons avec impatience et qui doit être dans cet amendement finalisé d'ici 2027. Voilà. Les 308 aussi, vous l'avez fait. Dans la foulée. Le 308. Il concerne effectivement 2 appels d'offres qui sont lancés par la DGA sur des munitions télé-opérées. Selon des méthodes effectivement extrêmement innovante est extrêmement intéressante. L'objectif ici et donc en présentant cette ces sous-amendements. Que ces munitions soit démission qui soit à bas coût. On a tous conscience aussi aujourd'hui de la nécessité d'avoir du volume et Damas et mais surtout du bas coût. Donc l'idée c'est vraiment que le coût unitaire de ce matériel ne dépasse pas 20.000 euros et donc le le sous-amendement précise que CMT devant. À Bakou

notamment le dispositif. J'ai j'ai AS. Pour soutenir la filière donc. À voir. Qu'on vient de renforcer la structuration de la filière des drônes et robots d'une part, cela permet de soutenir la BITD et les entreprises concernées. D'autre part, cette structuration facilite la protection des Start-Up et des entreprises de taille intermédiaire de robotique compte les tentatives de rachat des fonds d'investissements étrangers. Je ne cite pas les pays mais vous avez tous deviné comme l'a rappelé le rapport d'information dont je faisais référence tout à l'heure. Ne passons ensuite suite à l'amendement 89 de monsieur tu es mal. Merci madame présidente. Il s'agit là des systèmes d'armes létaux autonomes, donc les armes autonomes. Vous savez que les États-Unis, la Chine décide d'aller très loin et donc cet amendement vise à ce que la France promeut un un traité un accord multilatéral. Pour encadrer l'élaboration l'utilisation de ces armes-là parce que c'est un sujet pour le coup stratégique. Monsieur le Ministre et je crois qu'il est important qu'on porte sur cette voie là sur la question des armes autonomes. pour le 143. Hein madame Gréaume pardon. Si la France se doit effectivement protéger ses armées l'usage d'éventuels de tels systèmes. Les tout comme mon collègue vient de parler ne devrait être effectué que dans la plus grande transparence possible et sous le contrôle démocratique du Parlement cet amendement vise donc à soumettre. Le développement de ces systèmes à un débat devant le Parlement sur plusieurs points, notamment les incertitudes techniques et juridiques qui ne peuvent être pris à la légère. De plus, cet amendement visait également à ce que la France s'engage à accélérer les négociations diplomatiques autour de l'interdiction des systèmes d'armes les îles Merci, monsieur le Président vont tard pour le 221. Merci madame, madame la présidente. Nous comprenons que l'utilisation des drone s'inscrit dans le cadre de l'innovation technologique en matière de défense du plaisante sert des avantages technologiques majeures, il offre une capacité de surveillance et de reconnaissance sans précédent, ce qui permet aux forces militaires d'obtenir des renseignements précieux sur le Champ de bataille sans exposer directement les soldats des risques. Les drônes armés peuvent mener des frappes ciblées, minimisant ainsi les dommages collatéraux et les pertes humaines. Ils sont extrêmement mobiles et peuvent être déployées rapidement dans des zones d'intérêt, il pose des questions éthiques et juridiques majeurs et peuvent par exemple conduire à la violation de la souveraineté territoriale des États survoler ou être utilisées pour commettre des éliminations extrajudiciaires, rappelons que le droit international humanitaire interdit les armes qui ne permettent pas de respecter ces principes généraux nécessité distinction proportionnalité précaution et interdiction de causer des maux superflus. Or l'usage des drone dans des opérations militaires peut entraîner des violations des droits de l'homme en entraînant des victimes Simi civils et la surveillance exercée par les drônes soulève des préoccupations en matière de vie privée et de protection des données. Il est donc important de débats de ces questions éthiques et de mettre en place des quatre réglementaire des normes et des protocoles appropriés pour encadrer l'utilisation des drone militaire. Nous devons donc nous engager activement dans la recherche d'un équilibre entre l'efficacité opérationnelle et le respect des valeurs éthiques et du droit international humanitaire à l'échelle hein ah National. C'est pourquoi nous proposons que la France soit fer de lance de la construction d'un indispensable traité. International pour assurer un encadrement multilatéral de l'usage des drônes, armés ou d'espionnage. Merci Monsieur le Président quand bon quel est votre avis sur ces sous-amendements, amendements Pour l'amendement du gouvernement qui propose de réécrire le paragraphe sur les drônes et les robots c'est une réécriture qui comporte des compléments et des clarifications. Donc, la commission s'est prononcée favorablement. De même, la commission s'est prononcée favorablement sur les deux sous-amendements de nos collègues Perrin et Bono qui propose des sous-amendements utile à cet amendement du gouvernement d'une part pour accélérer l'armement du Patro leur bien sûr et pour que les munitions télé-opérées demeure à Bakou et ne soit pas sûr spécifiés ces sont les sous-amendement de notre collègue Cédric Perrin et bien sûr pour que la filière drone soient mieux structurer et accompagner notre collègue François Bonneau. ne ne l'avis de la commission est défavorable sur les trois amendements suivants 89 143 et 221 qui sont de toute façon incompatible avec la réécriture opérée par le gouvernement avec son amendement 274.

Qui s'abstient il est adopté le 89 ne tombe pas seul le 143 tombes. Voilà donc je vais mettre aux voix 89 qui a un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté de 143 est tombé et le 221 ne tombe et je mets aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Et nous passons maintenant à aux 40 de monsieur Oui madame la présidente. Monsieur le Ministre. Nous savons bien aujourd'hui notre pays ne sera pas confronté, dans l'avenir. Qui a des cons qui a des conflits asymétriques et donc nous devons nous préparer. À cette menace et et dans ce sens. L'artillerie sol-air devraient être développé amplifié pour l'avenir. Donc cet amendement qui est très simple VISA insister sur l'actualité des moyens de défense sol-air et leur prédominance ce sera. Belgique. Qui doit être amplifié. C'est un avis favorable sur un amendement qui du reste tient compte dans un rapport dans le rapport annexé du retour d'expérience des conflits tels que celui du Haut Karabach ou de l'Ukraine. Monsieur le Ministre votre avis oui favorable. Je mets aux voix de Baby favorable pied pour qui est contre qui s'abstient adopté le 2 75, monsieur. Monsieur le Ministre. Avis de Avis de la commission favorable je mets aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adopté le 26 monsieur Merci. La présidente. Cet amendement a pour objet d'essayer de trouver des solutions en matière de de base aérienne. Concernant la possibilité de les utiliser de façon duale entre une une activité civile et une activité militaire. Avis de la commission. Avis favorable à un président. Avis du ministre-défavorable je mais aux voix avis favorable de la commission défavorable du gouvernement. Et pour. Qui est contre ou, Qui s'abstient. On recommence, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le vent. Monsieur Sécurité, allez-y. C'est à vous.

Merci ben présidente. Cet amendement de notre collègue. Folio effectivement a pour objet d'essayer, comme l'a évoqué, Monsieur le Ministre précédemment de trouver une répartition prioritaire. En outre-mer pour des nouveaux moyens de projection sans précision aucune. Commission souhaitent demander l'avis du gouvernement sur cet amendement. que pour la. C'est la première loi de programmation militaire depuis pour le coup qu'elles existent dans lequel il y a autant de déclinaisons. D'ambition sur l'outre-mer. Après je veux bien construire dans un signalement pur dans lequel on on prend tous les, toutes les lignes et on y remet le mot outre-mer de là où je viens de mes fonctions ministérielles précédentes. Ce n'est pas pour me déplaire dans, donc pour des raisons de pure forme, j'ai mis un avis défavorable sur sur tous ces amendements parce qu'en fait on vient alourdir la copie pour quelque chose qui est déjà intégré par ailleurs Après avoir entendu l'avis du gouvernement. Quel est le vôtre, monsieur rapporteur président défavorable. Donc je mais aux voit double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 31. Oui et madame la présidente, monsieur le ministre. Cet amendement vise à proposer une concrétisation de la programmation militaire pour la souveraine souveraineté en outre-mer en formulant des nécessité de prépositionnés au moins frégates de premier rang par zone stratégique d'intérêt majeur en particulier dans l'indopacifique dans le but de consacrer à l'horizon 2030 les capacités nécessaires en termes de navires et d'infrastructures. Il nous faut en effet dès à présent organiser les capacités portuaires d'accueil en identifiant les zones susceptibles d'accueillir ces nouveaux moyens. C'est l'objet de cet amendement. quel est l'avis de la commission. Position de retrait sinon avis défavorable. Monsieur le Ministre. Défavorable pour les raisons exprimées président. Vous maintenez. Oui. Retirer.

Oui merci c'est un mot qui consiste à. Au moment où nous parlons de la politique cyber insérer le mot Sibérie et numérique dans notre stratégie. Parce que toute la politique cyber qui est annoncé dans le. Sel par le gouvernement dans dans dans ce. Dans cette loi de programmation militaire elle prétend assurer notre souveraineté en tout cas notre défense nos capacités offensives ou d'influence en matière cyber mais elle ne se préoccupe pas. Des couches intermédiaires du numérique. La production de logiciels de système d'exploitation. Les, les réseaux, les matériels les infrastructures réseaux et les composants électroniques, les matériels. Donc nous avons un problème on amont de souveraineté numérique majeur. et c'est pour ça que nous proposons de rajouter ça dont le titre ce sera complété par un amendement qui va suivre. Qui. Va dont donc dans le sens des compléments nécessaires à cette stratégie. La commission. Rédactionnelle avis favorable. Monsieur le Ministre. Défavorable défavorable. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Monsieur Bono le 47. Ah poursuivent hé bien accroître les moyens en la matière, qu'il s'agit d'un sujet. Indispensable en la matière. Quel est l'avis de la commission. C'est un amendement rédactionnel qui est satisfait par la l'actuelle rédaction du rapport annexé. Je propose de retirer cet amendement sinon l'avis est défavorable. Monsieur le ministre. la même chose que le président Cambon c'est déjà satisfait donc je disais mais c'est pas grave si c'est adopté donc favorable mais enfin donc. Retrait. Monsieur Bono, que faites-vous de tout ça.

a indiqué la la vulnérabilité des collectivités locales et territoriales au niveau cyber et d'ailleurs je peux témoigner de d'exemples assez précis en la matière. Souvent victimes d'attaques ou peu protéger. Ainsi que nos hôpitaux, nos mairies et services essentiels. Donc en ce sens, soutien appuyé, pourrait conduire à un accompagnement et une cellule de défense, le cas échéant par rapport à des attaques de type violente et étrangères Nathalie. Oui c'est un amendement qui. Qui vise à souligner le nécessaire effort de protection cyber des collectivités territoriales et des services publics qui avait à travers l'appui du ministère des Armées à l'Agence à Lancy, à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est important quand même de rappeler que cet appui au secteur civil par la cyber défense désormais ne s'entend bien évidemment qu'en cas de crise. L'Inde s'il doit rester l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales, avis favorable. l'enfer est pavé de bonnes intentions, ce que je vois très bien ce que vous voulez faire. Donc il y a pas de sujet sur le fond au global. Après dans ce paragraphe, là on est véritablement sur la cyberdéfense mises en oeuvre par le ministère des Armées. Dans le cas de la programmation militaire quand on parle de cyber désarmé. C'est pas d'Annecy. On est sur. EMA et DGSE et que pour le coup n'ont aucun lien avec les collectivités territoriales et si c'est l'accompagnement de l'Annecy au quotidien des collectivités. On est sur l'interministériel. On n'est pas sur le rapport annexé de la LPM, je. Sur le fond plutôt demande de retrait puisque la référence aux collectivités territoriales ici me semble pas au final la droite. Si on relit le texte a froid. Est-ce que vous retirez vous maintenez. Vous le maintenez donc cet amendement a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

on perd aussi en capacité donc il voulait à tu et à attirer l'attention. D'où l'ajout de la phrase qu'il propose Oui comme je l'ai dit précise précédemment la la l'efficacité d'une politique cyber en matière de défense, elle suppose la souveraineté numérique qui nous fait aujourd'hui profondément défaut. À nous d'ailleurs et à l'Europe en général. Il faut donc s'occuper de la question des matériels dont la conception et la fabrication. Nécessite l'euro développement de capacités nationales et européennes. Les États-Unis ont décidé de mener la guerre économique et technologique contre la Chine avec le Chips acte mais ils embarquent les Européens dans des partenariats qui nous inclus dans cette guerre économique. Je pense notamment à l'accord entre STMicroelectronics et GlobalFoundries en juillet dernier. Sur ce sujet. Or nous devrions plutôt chercher à sortir de cette dépendance à l'égard de la Chine. Évidemment, mais aussi à l'égard des États-Unis. Par ailleurs, notre dépendance en matière de logiciels, que ce soit à travers le système d'exploitation de nos ordinateurs ou les plateformes d'accès. N'est pas durablement tenable. Si nous ne voulons pas construire notre politique cyber sur du sable. Donc il faut s'occuper, évidemment. De contrôler les données les contenus mais il faut s'occuper du contenant et là aussi. Il y a défaut de politique industrielle, nous devrions donc réorganiser. Le travail pour une filière. National et les coopérations européennes de souveraineté en la matière et c'est le sens des. De l'amendement que nous proposons en complément de l'ajout du terme numérique à côté. Du terme cyber que nous avons adoptées précédemment. Oui, cet amendement barre d'une bonne intention en souhaitant que la France s'engage évidemment dans la à maîtriser la production de ses composants électroniques et l'ensemble de la chaîne numérique logiciel et d'infrastructures. Néanmoins il nous apparaît que. C'est une dimension européenne qu'il faut porter à cette ambition et c'est une ambition qui n'est pas singulièrement les moyens d'un seul pays. C'est ainsi par exemple que la la production, la production de puces électroniques les plus sophistiqués s'appuie sur une entreprise néerlandaise. C'est pourquoi la France ne nous paraît pas devoir et. Décider seul décideur et s'engager dans une stratégie C'est pour ça qu'on a préféré retenir l'amendement du gouvernement 268 qui a déjà été adoptée et dont la rédaction respecte l'environnement européen de la labellisation des solutions d'hébergement des données de confiance autrement appelé Claude ou info nuages. Ou avis défavorable. Même avis madame la présidente. Bien monsieur Laurent, vous maintenez. Donc double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté madame Conway Mouret le 185. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre. Les autres opérations d'armement forment l'épaisseur des forces des 3 armées et revêtent une importance majeure pour la cohérence capacitaire d'ensemble l'ont été au coeur de la précédente loi de programmation militaire qui avait été érigé à hauteur d'hommes et de femmes qui avaient été ajoutées au Sénat par. Un grand nombre d'amendements adoptés suite d'ailleurs au travail assez important qui avait été. Réalisé Réalisé à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances. Un rapport que je vous invite à consulter d'ailleurs par rapport au, au débat que nous avons eu hier les autres d'opérations d'armement sont toutefois moins visibles dans ce texte que les programmes à effet majeur cet amendement propose donc de faire apparaître quelques-uns des petits programmes nécessaires aux forces spéciales dans le rapport annexé. Favorable. Après le don de matériel à l'Ukraine, notamment dans le cas de la frappe de la prof dans la profondeur des fameux lance-roquettes unitaires Les et les rues. Il est évidemment nécessaire de procéder à la à la renouvellement de cette capacité, cette capacité pourrait potentiellement être j'allais dire couverte par une offre souveraine de d'entreprises françaises et cet amendement. Vise à garantir que cette solution de remplacement de lance-roquettes unitaires soit une solution qui soit effectivement souveraine qui intégrerait une capacité de frappe précise dans la profondeur par des missiles hypervéloces et intégrant et si le fait que, il faut évidemment le le au maximum chercher. La profondeur et la distance donc voilà le, l'objectif de cet amendement. Merci de la commission. Il est favorable à une solution souveraine, monsieur le ministre. On y est favorable. Et le plus vite possible et la question c'est quand, voilà c'est une conversation évidemment enfin l'amendement du sénateur Perrin fait suite. À une réunion de travail sur site. Si je veux dire qu'on a eu dans dans le régiment de son territoire. À Belfort. Enfin dans le Territoire de Belfort. Le sujet le suivant. Juste pour éclairer le Sénat en un mot et les rues. Châssis américain adaptation française accessoirement il y a le sujet, lire Ukraine mais même sans le sujet Ukraine quid des frappes en profondeur et de longue portée à l'avenir. Donc évidemment il y a pas de raison que ce segments échappe à notre réflexion souveraineté autonomie stratégique. Donc on a envie de le faire donc on mobilise notre BITD différentes entreprises que Shilpa qui peuvent évidemment ils répondent favorablement après il y a un quid opérationnel et d'ailleurs les les noter. Rien. Que nous étions en contact. On leur a posé la question, c'est entre une solution souveraine dans longtemps ou une solution mixte parce qu'elle serait jamais complètement étrangères enfin en tout cas comme le les rues faut regarder à plus court terme, il y a un débat au sein des armées. moi je veux le redire comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale toute solution souveraine sera toujours celle qu'on retiendra après il y a l'incertitude désormais évidemment du délai. Un peu aussi des coûts coûts normal faut aussi Challenge et l'industrie pour qu'on sorte une solution souveraine qui soit le plus adapté et sur le terrain opérationnel, la qualité du matériel mais aussi évidemment sur la soutenabilité pour le contribuable, ça je pense qu'on est tous d'accord avec ça

c'est comme ça qu'il faut comprendre l'amendement et je voulais juste le redire si vous 7h Perrin et d'accord sous cette réserve sagesse. Je ne dis pas favorable même si je suis d'accord avec le fond mais ça veut dire que tout doit être fait pour le faire dans la sincérité de la programmation.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement travailler avec Icahn France le relais national de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires vise à rappeler le plein respect du traité de Lisbonne et éviter toutes mes interprétations de l'alinéa 99 du rapport annexé de la LPM. La clause de défense mutuelle de l'article 42 7 du traité de Lisbonne de 2007 stipule bien que la défense des autres États membres de l'Union européenne en cas d'agression armée n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité de défense de certains États membres. Cette dernière phrase fait notamment référence à l'impossibilité pour la France d'user de ses armes de dissuasion nucléaire dans un tel contexte, les États de l'Union européenne ont en effet des États de l'Union européenne ont en effet ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires en l'occurrence. L'Autriche et l'Irlande qui stipule à l'article 1, que chaque État partie s'engage à ne jamais en aucune circonstance employer ni menacé d'employer des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires. Nous voulons donc par cet amendement, nous assurer que la France respecte bien ses engagements européens. Sur ce point précis. Merci. Alors. Cet amendement est évidemment satisfait puisque la dissuasion. La dissuasion française ne trouvent bien évidemment à s'appliquer qu'en cas de menace sur nos intérêts vitaux et donc il ne s'agit en aucun cas d'un quelconque parapluie nucléaire français. Dont pourrait bénéficier à un autre pays de l'Union européenne. Donc soit cet amendement est retiré sinon un avis défavorable. Monsieur le Ministre, oui mais la présence non non seulement défavorable. Si j'étais taquin, je dirais aussi que les les mêmes pays qui sont engagés dans les démarches du sont ceux qui sont à l'OTAN dans la planification nucléaire lorsqu'ils n'accueillent pas des bombes américaines sur leur sol. Donc c'est quand même toutes les limites aussi de cet exercice. Et que donc, au fond, notre modèle il est-ce qu'il est mais au moins il est cohérent, il est sincère et moi c'est ce que je redis un certain nombre de d'homologue de pays européens qui d'un côté pour satisfaire leur parlement ou des problèmes de coalition politique domestique s'engage sur le tien. Mais ensuite se précipitent pour intégrer les planification nucléaire de l'OTAN. Sous le parapluie nucléaire américain je pense que cette incohérence, là elle est désormais problématique pour beaucoup de partenaires européens puisqu'elle ne l'est pour nous même à bien des égards donc demande de retrait ou défavorable. Je mets aux voix double avis défavorable qui pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté Monsieur Gontard le 223. Merci madame la la présidente. Cet amendement vise à à donner une nouvelle impulsion politique étrangère collective de l'Union européenne. Nous sommes favorables à une Europe de la défense et nous pensons qu'elle doit être au coeur de nos débats sur notre modèle d'armée des coopérations et des mutualisations à l'échelle européenne nous permettrait d'avoir un modèle d'armée bien différente de l'actuelle cependant une Europe de la défense est complètement indissociable d'une politique étrangère européenne aujourd'hui cette nouvelle politique étrangère européenne est plus que jamais nécessaire. La guerre aux portes de l'Europe marque un moment charnière de l'Union Européenne et nous impose de rebâtir une politique étrangère collective. Cette politique étrangère commune, permettrait à l'Union européenne de parler au maximum d'une seule et même voix en prenant des positions fortes et unifiée sur les questions internationales cette unification nous permettra de gagner en crédibilité en autorité auprès des autres acteurs mondiaux, ce qui est un élément stratégique non négligeable. Nous serions alors plus actif et plus efficace dans plusieurs secteurs, comme la résolution des conflits. La promotion de la démocratie et des droits de l'homme et la gestion des crises humanitaires. Alors que les décennies qui viennent, seront marqués par un affrontement de bloc entre les superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. La seule manière pour les pays européens de faire entendre leur voix dans le concert des nations et de les harmoniser pour n'en avoir qu'une. ambitieuse. L'Union européenne, donc on donne un avis Forum favorable même si cet amendement est un peu limite, par rapport à l'objet de la loi de programmation militaire. Monsieur le Ministre. suite de la phrase comme cet amendement est très éloigné de ce qu'est la programmation militaire même si sur le fond ne présente pas de difficultés, avis défavorable, parce que à la fin on va avoir un rapport annexé quand même qui va plus ressembler à grand chose par non mais c'est pas du mépris par rapport au fond de ce que vous portez. Mais si on est sûr rapport annexé une programmation militaire. Il faut être honnête, là on s'éloigne quand même fortement de l'affaire. C'est c'est c'est

Oui, c'est un moment d'appel. Ce que nous souhaitons a au très haut, cet amendement avant la position du gouvernement sur le projet sur les négociations sur l'accord ASAP. Donc c'était plutôt pour avoir cette discussion-là certes rapidement à l'heure où nous sommes. Mais il nous semble important d'entendre au moins la position du gouvernement. Très bien, j'ai quand même solliciter l'avis de la commission. La Commission pense qu'il conviendrait d'attente que la négociation soit stabilisé, d'autant que cette négociation est particulièrement complexe et mouvementée et elle pose de vraies questions sur le fond. La vie la commission était défavorable. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, alors j'il y a le fond de l'amendement et à ça parce qu'on est un peu éloignée. Le fond de l'amendement quand même et d'intéressant. Demande de retrait pour celui-ci, sur le fond. Faut-il imaginer un commandement européen en plus du commandement intégré c'était le le contenu de l'amendement en tant que telle. Alors la réponse est non. Faut-il en revanche avoir au sein de l'OTAN et là ça permet quand même de rebondir si veut. DG parce qu'on n'a pas eu le temps de parler suffisamment de l'Alliance Atlantique. Est-ce que il faut que le pilier européen de l'OTAN, si on reprend les terminologies. Retenue doit être plus fort. La réponse est oui et pour ça il est évident qu'il faut que la France au sein de l'OTAN soit beaucoup plus forte qu'elle ne l'est. Alors comment peut-elle être j'ai largement parlé des 2% du PIB. Je reviens pas mais j'à travers ASAP parce que ça pose la question de ou est-ce que là où le contribuable européen, mais de l'argent pour se réarmer. Comment ça profite à la BITD eux et donc à notre autonomie stratégique européenne et donc je sais que ce soir d'ailleurs à l'emploi européen parce que même si c'est fait pour se défendent de produire des armes, il y a aussi quand même un enjeu de de de capter de fixer la production de richesses. Des dépenses militaires sur le, sur le territoire européen ce j'en dirai un mot dans un instant, 2% du PIB. Je reviens pas commandement intégré. De fait, monsieur le sénateur, c'est mal, il faut qu'on soit moteur. Nous le sommes parce que comme on a un gros contributeur militaire. Je rappelle au Sénat. Chaque année, chaque pays membre de l'Alliance c'est une. Promesse de mise à disposition de moyens militaires, donc ça c'est pour ça que je j'étais dur sur les 2% parce que c'est la différence entre avoir du matériel dans un hangar et de dire, je mets un nombre de bateaux un nombre d'avions, le cas échéant des troupes au sol à à la disposition de de sa heures du commandement intégré sur lequel je le dis tout de suite. Pour certaines sensibilités politiques, nous gardons le contrôle national de ce que font les forces. forces. Important parce que souvent dans les critiques sur le commandement intégré de l'impression que c'est Washington qui devient. Le le le commandement suprême des forces françaises qui sont versées au pot du gouvernement intégré, certains pays, peut être le fond. fond. Ce n'est pas du tout. Bah, je suis désolé, demander au chef d'État-Major des armées, lorsque vous l'auditionner. En en commission, vous avez et moi d'ailleurs je le vois passer au quotidien comme Ministre vous avez toujours un contrôle national. Des forces qui sont versées l'OTAN toujours et ça pour le coup c'est notre constitution, ce serait anticonstitutionnel. De toute façon ça ne se passe pas. Donc première chose continuer, être exemplaire. Je ne veux pas être critique ou désobligeants. On a beaucoup de pays, y compris des pays voisins. Compris et des pays avec lequel on a parfois des coopérations importantes. Qui font beaucoup de promesses de mise à disposition de moyens militaires et qui derrière dans l'exécution ne le font pas, nous on fait partie des deux premiers pays de l'Alliance dans lequel ce qui est promis est vraiment mis à disposition ce qui fait que sur le terrain militaire, on est plutôt crédible dans le commandement intégré 3ème des choses, il y a un combat à mener. Sur les civils au sein de l'OTAN. Alors il y a même. Amener n'est pas là mais il y a évidemment l'Assemblée parlementaire. De l'OTAN. Il y a évidemment les postes civils au sein de l'OTAN. Qui est pour moi un point clé de la discussion avec le secrétaire général de l'OTAN. Nous avions. Jusqu'à peu un secrétaire général adjoint, ou en tout cas l'équivalent de 2 délégués. Qui. Et Camille Grand. Il n'a pas été remplacée par un français, donc ça c'est un point de vigilance sur lequel, je pense qu'il faut qu'on soit évidemment évidemment très allant. Et puis il y a là il y a la réactivité. Monsieur le sénateur es mal lorsque on fait Roumanie ou police du ciel en Estonie ou en Pologne. Il est clair que pour le coup, on est véritablement dans le temps militaire très concret pardon de ce dégagement, un peu long mais on a on va. Prendre le dernier virage avant la les 30 amendements qui reste et on a pratiquement pas parlé d'autant. Donc je voulais redire quand même que on ne peut pas comprendre la loi de programmation militaire. Si on ne l'armée pas dans le cadre de ses alliances et et ça c'est absolument clé compris pour le format d'armée c'était la conversation que nous avions avec les, les élus communistes de l'Assemblée, comme du Sénat. Il est clair qu'au moment enfin autant ou pas autant et dissuasion nucléaire ou pas. Dissuasion nucléaire, ça ne fait pas le même format pour l'armée de terre, ça ne fait pas le même format pour l'armée de l'air et ça ne fait pas le même format pour la marine, ça c'est une réalité. Ensuite ASAP. Initiative de Thierry Breton comme commissaire. Européen qui, au fond, comparaison n'est pas raison mais de se dire, il s'est passé suffisamment de choses sur les vaccins pendant le Covid pour qu'on ne se pose pas la même question sur l'équipement militaire au moment où il faut aider l'Ukraine. Je le fais vite mais enfin globalement le raisonnement et et celui-ci. Là pour le coup, Thierry Breton actionner plusieurs leviers alors qu'ils viennent aussi reprend l'agenda de Versailles qu'on avait commencé à dessiner. Et Dieppe et dire pas les capacités à acheter en commun les instruments de financement commun le Fed le Fonds européen de défense dont d'ailleurs la France bénéficie d'un d'un bon retour sur ASAP les, les discussions sont toujours en cours au Parlement, Conseil Commission dans le trio, j'allais dire infernal. En tout cas. Le trio telle que prévue par les traités. Et ce pour lequel nous on est très allant sur le dispositif avec les éternels ligne rouge française que vous connaissez, que je vous partagez c'est évidemment attention sur la doctrine d'exportation d'armes de la France, il s'agit pas de communautariser elle doit rester nationale enfin je je veux pas tous les citer mais vous les, vous les connaissez par ailleurs en tout cas c'est clés. Je pense aussi que ces clés dans l'acceptabilité de des dépenses publiques militaire. Et on revient aux 2% du PIB, ce qui avait été dit d'ailleurs par le président Laurent c'est que au bout d'un moment quand même, c'est de l'argent du contribuable européen. Il faut que ça profite à l'industrie européenne et si possible française dans cette affaire et pas l'industrie américaine. Je crois que c'est quelque chose qui ont tant entendu pour nous vous autres Français sur lequel on peut se rejoindre, en tout cas, ça mérite d'être, d'être accompagnés. Si Thierry Breton arrive emmener le paquet jusqu'au bout qu'on le veuille ou non ça sera un vrai virage dans l'Europe de la défense, il sera peut-être pas spectaculaire parce que moins symbolique à l'abri la brigade franco-allemande. Mais si on y regarde de près, il fera certainement plus efficace plus durable et plus transformant et en fait je crois que l'Ukraine nous oblige à nous poser les bonnes questions sur la coordination entre Européens qui au fond revient aussi à des coordinations sur le volet industriel sur le volet Marché commun sur ces sujets sur lequel en plus nous autres Français, on a la BITD qui nous permettra en plus d'air, d'aller chercher, à mon avis quelques promesses à l'export en Europe. en Europe. Dans ce cas de configuration là je pense très fort aussi au sujet des munitions. Voilà, de manière un peu longue pardon mais au moins je vous aurais répondu à votre DG auquel je n'avais pas répondu. Depuis 3 jours. Monsieur tu es mal vous voulez retirer votre amendement j'imagine.

Madame la présidente. Merci. En fait, Monsieur le Ministre, cet amendement s'inscrit parfaitement dans ce que vous venez de développer, c'est-à-dire votre volonté finalement de de renforcer et de consolider la BITD Nous partageons la même ambition européenne. Que l'on peut trouver dans le discours de de l'exécutif et et nous avons pensé qu'il était nécessaire de réaffirmer cette volonté en fait dans le rapport annexé. D'abord parce que elle est historiquement lié à ce que nous avons toujours défendu mais aussi parce qu'aujourd'hui, le contexte international, finalement nous oblige à nous unir. Je crois que nous avons traversé une série de de crises successives qui font que nous avons une opportunité. Peut-être unique de consolider l'Europe des 27 et notre singularité stratégique ne doit pas nous empêcher de nous tourner vers nos partenaires européens pour établir des coopérations de défense mais aussi pour pouvoir exporter nos matériels sont quoi. Nos partenaires européens s'organiseront autrement sans nous et nous en avons déjà malheureusement. Quelques prémices.

Si on nous avait dit il y a quelques années qu'on était capable d'avoir un fonds mutualistes. Avec un système de remboursement qui permet d'aider à la fois des pays d'Afrique mais aussi désormais essentiellement l'Ukraine. C'est le quand même l'Europe de la défense de manière très concrète, je voulais quand même le signaler. Non sur l'amendement favorable. Ça porte un mot aussi hein c'est le nom d'une entreprise, c'est par exemple MBDA c'est qu'on voit bien aussi que désormais on a des entreprises qui sont compatibles avec notre souveraineté dont l'organisation interne, d'ailleurs, correspond aussi à un partage. Souverain je dirais MBDA. Grande-Bretagne Médéa Italie MBDA France les règles du jeu sont sont absolument connue et et clés et en même temps ça nous fait un champion européen le vrai. La vraie question et je le pose ici comme réflexion pour l'avenir, c'est quels sont les autres modèles de cette nature que l'on peut envisager sur d'autres segments capacitaire pour nous permettre aussi d'être solide 3ème point partenariat européen alors 1000 fois oui mais j'ouvre. On a aussi une vocation indopacifique. Donc tout ce qu'on fait en européens se fait en plus de ce que l'on peut faire avec, Émirats Arabes Unis, Inde, Indonésie, que sais-je. En tout cas a aussi cette vocation là et donc au fond, notre identité, c'est d'arriver à marcher sur ses 2 jambes.

Dans les textes autonomie stratégique européenne. Toutes les lignes mais toutes les décisions qui ont été prises. Depuis le début de la guerre en Ukraine nous éloigne de cette perspective. Déjà le débat était très compliqué au moment à où il était question de simplement écrire à la formule autonomie stratégique européenne dans les documents d'orientation de l'Europe, sur ces, ces questions mais. Nous avançons à à l'opposé, à l'opposé de cela la remilitarisation de l'Europe, comme je le disais. Hier, elle se fait au profit des industries d'armement américaines en très grande partie nous donnons dégage. Vous nous avons laissé faire. Ah les les l'adhésion de la Suède et de la Finlande sous la enfin ça va peut-être se terminer à Vilnius. On verra sous la presse sous le chantage des de la Turquie. On laisse en faire hein et en obligeant ces pays a signé un mémorandum avec la Turquie sur les conditions de leur adhésion. lauriers à des pays à des régimes politiques de l'Est européen. A qui quand même sont très éloignées. De conceptions démocratique. tout ça nous éloigne de cela, il faut quand même dire ça parce que après on peut écrire. Autonomie stratégique européenne mais entre autonomie stratégique européenne et commandement intégré de l'OTAN. Je suis désolée parce que vous aviez révoqué ça Monsieur le Ministre. Il faudra un jour choisir. Mais les 2 ne sont pas compatibles et à force de dire que c'est compatible, hé bien en vérité nous ne traitons pas en profondeur et sérieusement le sujet d'une éventuelle. Construction d'une autonomie stratégique européenne. Alors je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis favorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté le 91 madame Gonod mourait. Oui madame la présidente. Monsieur le Ministre, en fait, cet amendement vise à permettre à chaque ambassade de disposer d'un attaché de de défense alors c'est pas simplement parce que nous en avons besoin pour nous avons besoin de sa présence pardon. Pour organiser les JDC. Nous avons eu ce débat hier mais. Mais notre ambition et et finalement de de fabriquer pour pour exporter le no certains grands groupes hé bien les exportations représentent jusqu'à 60% du chiffre d'affaires et donc la présence, en permanence d'un attaché défense nous permettra d'abord de connaître attends les opportunités à venir de tisser des Liens avec les autorités locales et aussi de consolider des partenariats stratégiques qui sont essentiels à à l'achat de de matériel, pas forcément toujours pour le leur qualité mais en tout cas pour le lien que cela. Entre l'acheteur et le vendeur. C'est un avis très favorable sur un amendement qui est important et qui reprend. Ce que la commission des Affaires étrangères et de la Défense a souvent rappelé en effet cet amendement qui vise à doter d'un attaché de défense tous les pays alliés de la France ou membre de l'OTAN. Prend certes acte du fait que nous avons actuellement 90 attaché militaire de défense, couvrant quelque 165 pays dans le monde, alors bien sûr avec nos alliés traditionnels mais aussi l'Égypte. Les Émirats arabes unis, l'Inde, mais on va bien au-delà. Oman, Ouganda, Afrique du Sud, Chine bénéficie d'un un attaché de N'attaché de défense à l'inverse est étrangement certains pays membres de l'OTAN ne dispose pas de cet attaché de défense résidents. C'est le cas de la Léttonie de la Bulgarie, la Slovaquie, de la Slovénie notamment ils sont couverts par un autre chargé de défense et à chaque fois que nous rencontrons, ses dirigeants. ils émettent le voeu qu'un attaché de défense résidant. Leur soit désigné et donc nous nous sommes émus à plusieurs reprises de cette situation. votre. De de vous Monsieur le Ministre, une réponse et j'allais presque dire un engagement de votre part parce que ce sont des alliés fidèles dans lequel du reste nous avons. Même en Léttonie. Nous avons aussi les troupes. De manière alternative avec les 2 autres pays baltes, donc je pense qu'il serait important d'avoir là un attaché militaire résidents. Quel est votre avis. Monsieur le Ministre. Oui je. M'Ministre je disais déjà exprimé en commission est en train de, en train de remédier à ça. De plusieurs manières. Déjà de manière large dans certains pays on a un sujet non pas attaché de défense mains tachées d'armement. Lors du débat en Afrique moi je rouvre le du sujet global pour le comprendre parce que c'est une manoeuvre d'égérie. Au complet. Et donc moi j'ai souhaité typiquement pour le continent africain sur une liste de pays précis avoir un officier général de la DGA comme attaché d'armement, donc ça c'est un 1er point c'est parfois un besoin qui est plus précis qui attaché de défense. 2ème des choses, vous avez des endroits dans lequel il y a attaché de défense résidents ou non résidents. Ça, c'est évidemment un sujet que je suis en train de réouvrir puisqu'en fonction de l'évolution des partenariats. Dans un certain nombre de cas de figure, ça vaut le coup et. Pour être dans d'autres pays au regard de la relation de défense avoir un officier supérieur à plein temps. La question peut se poser. Donc ça, moi j'ai demandé une petite étude un peu flash sur cette affaire pour évidemment regardée 3 sur l'amendement en question sur le principe c'est oui après ce que l'Estonie et Malte ont vocation à être traités de la même manière entre résidents et non-résidents. On voit bien que non mais sur les pays baltes pour ne prendre que cet exemple là au regard de ce qui est actuellement en cours réassurance du flanc oriental. Évidemment ils sont à la frontière avec qui vous savez et cetera, ça vaut évidemment le coup de de muscler donc. Avis, avis favorable. Et au-delà de ça, je reviendrai devant la commission pour dire comment cette affaire justement trouvera son exécution. Merci je mets aux voix double avis favorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Ensuite nous avons un 100. Toujours Madame quand Dernier amendement sur l'Europe. La gare de l'Ukraine a déplacé le centre de gravité du continent vers l'Est élargit la vision d'une Europe centrée sur son noyau dur, composé des membres historiques à une Europe plus inclusive. Les pays d'Europe centrale, orientale et du Nord se retrouve au coeur de la nouvelle donne géostratégique à titre d'exemple, la Pologne est aujourd'hui le 1er pays de l'UE en matière de soutien militaire à l'Ukraine et la Première ministre estonienne a lancé l'idée d'un mécanisme d'achat conjoint de munitions au Conseil européen du 9 février dernier nous observer un véritable changement de paradigme. Suite au référendum. Le Danemark a récemment approuvé son adhésion à la politique de sécurité et de défense commune de l'UE, mettant fin à 30 ans de non participation du pays à la défense européenne. La Finlande et la Suède ont-elles mis fin à des décennies de neutralité en demandant à rejoindre l'OTAN, à l'image de la Pologne qui a annoncé son doublement de son. Budget militaire en 2023 pour atteindre 4% du PIB. L'ensemble des pays européens augmentent de manière inédite depuis des décennies leur budget de défense. Pardon, malheureusement à l'achat massif de matériel non européens. Comme il est fort probable que cet effort sera soutenue dans le temps, il serait opportun de saisir cette opportunité pour lancer des projets industriels en coopération avec le plus grand nombre de nos partenaires européens. Nous possédons déjà les outils à commencer par le Fonds européen de défense, cet amendement propose donc de prendre en compte cette évolution dans notre politique partenariale européenne par exemple nous pourrions rejoint l'Estonie, qui entend devenir un acteur majeur en cyber Space enfin cet amendement vise ainsi à élargir la liste des pays avec lesquels nous menons des projets capacitaire en coopération à l'ensemble de nos partenaires européens. Au-delà de nos partenaires historiques d'ores et déjà cité dans le texte. Monsieur le Ministre. Favorable, même la prise. Jamais aux voix doublées favorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adopté. À l'article 2 du rapport annexé, un amendement du gouvernement. Oui, mesdames, messieurs les sénateurs. En m'adressant directement au président Cambon sur cet Mans pour comprendre pourquoi on mais l'amendement du gouvernement. En fait moi je vois bien l'esprit je peux y souscrire. Le sujet c'est la l'interprétation. Je m'explique. À cet égard humeur articulations toutes les vérifications effectuées par la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre et celles opérées par les banques dans le cadre de leur contrôle de conformité sur à rechercher qu'est la crainte du gouvernement dans cette affaire, c'est de mettre. Sur le même pied d'égalité. Un contrôle réalisé par la et le contrôle réalisé par les banques enfin en aucun cas les banques un contrôle des banques ne pourra se substituer au seul contrôle qui vaille, à nos yeux évidemment celui de la Commission interministérielle. Je pense qu'on peut le comprendre, et accessoirement aussi monsieur le président pour la BITD, il ne faut pas que les banques refasse les mêmes procédures que ce que la sienne a déjà fait parce que là pour le coup, on va vers quelque chose qui peut un peu lourd. C'est l'esprit de l'amendement. Qui est pas de revenir sur tout ce que le Sénat a introduit en commission c'est juste là l'affaire. Telle que c'est écrit l'affaire Bank donne l'impression que le contrôle bancaire le contrôle de la scène se vaut. Il ne peut en être évidemment le le cas. Monsieur le Président, bon.

n'est pas d'affaiblir ce contrôle mais surtout d'éviter aux banques de mener des vérifications qui aurait déjà été opéré pas la siège alors peut-être il y a peut-être, on peut sous-amendé pour que soit bien compris car ça ça vise effectivement à simplifier les procédures administratives pour les entreprises de la BITD. Donc il y a pas du tout de volonté de contester. si ce n'est que l'écriture ne peut introduire évidemment ce ce cette confusion. Une meilleure articulation entre les vérifications effectuées. Je pense qu'il faut le dire comme vous venez de enfin faut l'écrire Le ministre comme il s'agit d'un amendement assez succinct dans sa rédaction et pardonnez-moi, laissez-moi finir. Et pour le sous-amendé. Je vous suggère de nous transmettre une rédaction à cet instant. Oui alors si on est complètement cohérent puisque c'est le Sénat qui a modifié le texte en commission, je pense que c'est bien que ce soit sur ce sujet. La commission qui amende pour être complètement transparent. Voilà ça fait donc suspendre quelques instants pour que la commission donne une rédaction.

Monsieur mise donner votre avis sur ce nouvel amendement de la commission et nous dire ce qu'il advient du vôtre. Retrait de l'amendement du gouvernement. À mon avis favorable du gouvernement sur l'amendement du président Voilà alors donc je mais aux voix ce nouvel amendement de la commission qui a un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Monsieur président Gontard. C'est à vous pour le 225. Oui merci madame la présidente. Nous souhaitons par cet amendement. Inspiré notamment par Amnesty International et les travaux du Parlement européen que la France respecte ses engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme et cesse l'exportation d'armes dans les pays autoritaires ou les droits de l'homme sont bafoués ou l'utilisation d'armes et détourné pour réprimer la population réduire à la perte des libertés civiles et commettre des abus graves. La France a vendu pour plus de 10 milliards d'euros de matériel militaire à l'Arabie ça doit en 2010 en 2010 et 2019 pour plus de 4 milliards aux Émirats arabes unis et pour plus de 7 milliards d'euros de matériel militaire à l'Égypte entre 2010 et 2019. Le média disclose a également révélé que l'État français a accordé 4040 licences d'exportation de biens à double usage en 2021 pour 9 milliards d'euros, avec pour principaux bénéficiaires. La Chine et la Russie. La surveillance massive de la population chinoise par le régime chinois et la répression dans le sang des Ouïgours nous a pas empêché de fournir au régime chinois des technologies de cybersurveillance. La guerre en Ukraine et les velléités impérialistes préalable de Poutine n'ont pas non plus interrompu de transfert de technologies liées au nucléaire civil. Les répressions sanglantes commises par les régimes égyptiens et libyens ne sont pas empêchés de leur fournir des technologies de surveillance. De surveillance de leur population contribue ainsi à ces violations des droits de l'homme en finançant entre autres la guerre au Yémen et la répression des populations par des régimes autoritaires n'est pas acceptable pour notre démocratie. La France doit respecter les articles 6 et 7 du traité sur le commerce des armes. Adopté à l'ONU en 2013. Respecter les règlements européens en la matière et réaffirmé son engagement en matière de droits de l'homme de stabilité régionale de paix mondiale de contrôle des armes et d'impact humanitaire. la commission rappelle que la procédure d'autorisation des exportations d'armement relève de la seule responsabilité de l'exécutif. En revanche, la question du contrôle parlementaire a posteriori des exportations est un sujet

de notre commission par. Pour la création d'une commission de vérification au sein de la DPR, ça a été longuement discuté hier. Donc je propose que cet amendement soit retiré. Par ailleurs, je me, je note que cet amendement mentionne très défavorablement des pays comme l'Égypte et les Émirats arabes unis, qui je le rappelle sont des partenaires stratégiques de la France, il faut quand même signaler que le repositionnement de la de de la France au Sahel a été rendu possible en partie grâce à l'aide apportée par les avions de transport des Émirats je tenais quand même à rappeler ce point je vous propose donc de retirer cet amendement. Monsieur le Ministre défavorable. Au collège. Donc je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Monsieur K. Merci madame la présidente. Dans son discours à l'école de guerre en février 2020, le président de la République, a affirmé l'impérieuse nécessité de l'indépendance technologique de l'Europe et sa capacité à anticiper les prochaines rupture stratégique. Il nous faut pour cela une BITD autonome et compétitive, un effort massif d'innovation la maîtrise de nos technologies de sécurité et la maîtrise de nos exportations de défense. Cela nécessite une politique industrielle des standards de souveraineté, car notre incapacité à penser ensemble nos intérêts souverains, mais chaque jour en cause notre crédibilité en tant qu'Européen, elle offre aux autres puissances, la possibilité de nous diviser, de nous affaiblir. En 2020 et 2022, la cession programmée des sociétés sensibles Photonis Excelya à des groupes industriels non-européens a plongé le gouvernement dans une situation très délicate. pas raison. Le modus operandi operandi du contrôle des investissements étrangers aux États-Unis c'est fille US permet le dialogue en amont pour définir les règles du jeu. Il s'agit ici de mettre en place de la veille et du contrôle a priori des investissements étrangers plutôt qu'à posteriori. Cet amendement va, va dans le sens d'une plus grande protection du savoir-faire des PME de l'industrie de défense française et attire l'attention du gouvernement. S'agissant des sessions de PME sensible de la BITD en permettant à la DGA. De limiter le Champ des candidatures, donc c'est un avis favorable. Ministre. Oui merci beaucoup madame la présidente. De fait, Célia le bon dossier de ce que nous sommes capables de faire et d'ailleurs moi je vous invite à. Peut être rencontré le le président d'Excelya. De voir comment les choses justement sont en en train de s'exécuter et qui au fond quand on voit la récupération politique de certains. D'une sensibilité qui n'est pas représenté ici au Sénat. Sur cette affaire, laissant penser au fond que tout était fait pour brader les intérêts du pays et cetera qui a été fait donc bon ça, ça montre bien que il y a pas de candeur, il y a la volonté politique et que il y a même des outils qui fonctionne bien. Première chose 2ème chose l'amendement et bon peut-être une demande de rectification toute simple, c'est de la DGA veillera en amont la DGA veille le tout veille le tout simplement au présent un présent prescriptif mais qui correspond aussi à ce que la DGA fait déjà. Et et je l'ai dit parce que. À l'Assemblée, je le refais ici je tiens vraiment c'est lui le l'engagement remarquable. Des équipes de la délégation générale pour l'armement du ministère en général parce que c'est eux qui font à la fois qui déclenche l'alerte, y compris pour Bercy qui la documente sur le terrain de la souveraineté ou le cas échéant la Direction des Applications Militaires quand ça touche à la dissuasion. Il y a vraiment un réflexe au sein du ministère des Armées avec des gens qui donnent beaucoup pour cette affaire. Et donc voilà. Juste une cette petite rectification et un avis favorable. Bienvenue. Mais ce Merci beaucoup monsieur le Ministre, effectivement je je l'ai vu aussi par exemple dans le dossier Photonis que j'ai suivi de vraiment de près. C'était déjà très avancée, effectivement le travail collectif et je voudrais dire que votre prédécesseur. A eu une action très forte pour éviter que justement Photonis partent

Alors il y a un sous-amendement enfin une rectification la rectification consiste à remplacer veillera par veille donc de passer du futur au présent. Dans le 1er verbe de la 2ème ligne. Tout le monde a. Intégrer donc je mais aux voix de vous êtes favorable pied pour qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Monsieur le président Gontard avec 226. Oui merci madame la présidente. Le programme Scaf et l'avenir de notre armée de l'air le système de combat aérien du futur n'est pas qu'un simple avion mais un système plus global avec des drone autonomes des avions ravitailleurs et avions de surveillance articulant notamment sur un avion de nouvelle génération furtif dit de 6ème génération cet avion sera doté d'armes novatrices tels que les drone et un dispositif connecté via le cloud de combat européen qui permettra à celui-ci d'être connectés en temps réel à d'autres avions comme le Rafale ou l'Eurofighter pour une utilisation des informations qui augmenterait la force de l'armée de l'air. Ce programme européen se décompose en plusieurs phases, particulièrement sur le NDF et sur les drônes comme dans toute démocratie parlementaire digne de ce nom ces phases sont outre-Rhin soumise au vote des parlementaires. Pour avoir un programme légitime aux yeux des Européens alors que notre commission ne cesse, à chaque occasion d'interroger le mini sur les évolutions du programme Scaf des débats et des votes sur les rapports de l'état de l'avancement du programme phase par phase permet également aux parlementaires d'être à jour sur le projet. Démocratiser la politique de défense en particulier lorsqu'elles impliquent des partenaires stratégiques, en y associant la représentation nationale, contribue à légitimer ces coopérations en leur conférant l'approbation de la représentation nationale, cela renforcerait également comme l'Allemagne, l'illustre à chaque sommet européen. La force de négociation de la France dans ses coopérations européennes. Il. Apparaît à la commission que la procédure. Est déjà assez complexe pour la mise en oeuvre de cette coopération qui naît se déroule pas sans difficulté. Nous ne sommes pas favorables à cette disposition qui vise à insérer la validation du Parlement à chaque nouvelle phase il nous apparaît en revanche qu'en application, je crois que c'est là l'article 108 du rapport annexé le gouvernement pourra faire une information du Parlement. Notamment. Les points d'étape lorsque on aura passé les travaux de la phase 1 B avant de passer à la phase 2 avis défavorable. Monsieur le Ministre. Oui, en fait, avis défavorable, parce que satisfait par cet équilibre qui avait été trouvé en discutant avec les différentes sensibilités politiques de l'Assemblée et du Sénat en disant que au bout d'un moment, ce sont des programmes importants avec beaucoup d'argent en jeu c'est bizarre entre chaque phase qui est pas une information au Parlement et mieux que cela. Moi j'ai souhaité que cette information est forcément lieu avant la loi de finances initiale de l'année qui enclenchera la phase suivante du SCAF. En clair, il y aura bien un vote du parlement, il se passera par ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire les crédits les abus et les CP en loi de finances. Donc ça c'était ce qui avait été trouvé. C'est ce que j'avais entendu en commission ici c'est ce que j'avais entendu en commission. À l'Assemblée nationale et c'est ce qui a donné lieu à ce qui a été introduit dans le texte à la demande de retrait au bénéfice de la rédaction qui a déjà été adopté par ailleurs. Il est retiré. Nous passons donc aux 281 du gouvernement. il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre ce que le rapport annexé doit donner comme indicateur. Pour permettre au Parlement de contrôler l'action du gouvernement et avoir des points de repère dans la programmation. Ça ça me semble évident. Même si ça pas toujours été le cas dans le programme en tout cas ça me semble être dans le bon sens. De. Un tableau qui prescrivaient de manière rigide. Des indicateurs qui s'imposeraient aux états majors venir c'est un peu la poule et l'oeuf notre affaire. Et donc ça pose la question du jalonnement des indicateurs alors en cela les demandes sur la disponibilité. c'est un exemple mais sur la disponibilité technique du matériel. C'était un des points attendus par la commission je suis engagé, je le redis ici même. Et donc j'ai déposé un amendement. Supplémentaire. Qui serait au fond un engagement du gouvernement. À ce que chaque année on présente au Parlement un bilan exhaustif. De l'activité de préparation opérationnelle des armées ainsi que le niveau disponibilité atteint par les matériels majeurs, je trouve que l'amendement de suppression, là c'est un moment de suppression de ce qu'elle fait la commission donc je peux comprendre que c'est un peu sec. Ça je l'entends bien et donc je, je veux faire cette contre-proposition voilà c'est pas un tableau qui prescrit déchiffrer égide vous états majors. Mais non en même temps dans la surveillance de la programmation. Il faut donc que le gouvernement viennent avec des données devant le Parlement pour pouvoir la contrôler. À discuter, mais en tout cas je je je j'accompagne donc les amendements de suppression qui vont venir du gouvernement par un amendement d'engagement du gouvernement dans la loi a donné un certain nombre d'indicateurs. S'il y a besoin. Je vous laisse le le cas échéant de regarder en tout cas c'est une présentation commune à l'ensemble des amendements madame la. Oui alors comme de toute façon, cet amendement ne vient pas à cet à cet endroit-là de la discussion. Ça va laisser un peu de temps à la Commission pour l'examiner. Voilà donc on le reprend et je sollicite juste votre avis sur le 280. Monsieur le Président quand bon. Alors compte tenu de l'engagement du gouvernement qui vient d'être exprimé pas par le ministre sur les informations. Que vous nous donnerez. Selon le format adapté qui a été souhaitée par nombre d'entre nous. Je donne un avis favorable à l'amendement du gouvernement et par voie de conséquence, je retire l'amendement 306 de la commission. OK. Je mais on voit cet amendement 280 du gouvernement avec avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Ensuite le 278. Monsieur le Ministre. Défendu sur la base du même argumentaire que précédemment évoqués. D'accord monsieur Bono. Le deux Oui madame la présidente. Tout étant important et. Non opposable par rapport par des questions budgétaires qui ont déjà été. Je je vais retirer cet amendement sachant que malgré tout, sur le plan terrestre le sujet existent. Quel est David la commission sur le 278 du gouvernement, avis favorable. Madame la présidente qui je mais aux voit qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Monsieur Perrin. 19. 19. La présidence. Monsieur le Ministre, le service de santé des armées assument une mission fondamentale en important à nos militaires. Qui acceptent de risquer leur vie au service de la nation, l'assurance d'être rapidement pris en charge et évacuer en cas de blessure. Le service de santé dans armées a pourtant vu ses moyens diminuer considérablement ces dernières années. Or la dégradation du contexte stratégique qui ont renforcé la probabilité d'un conflit de haute intensité, fait de la remontée en puissance du SSA un impératif absolu en particulier pour assurer sa capacité à gérer sur les théâtres d'opérations, un afflux important de blessés dans ce contexte le présent amendement vise à préciser que certaines capacités essentielles à cette fin, devront faire l'objet d'une attention particulière. On entend on étant réévaluer au cours de la période de la programmation et le cas échéant renforcée pour répondre aux besoins identifiés. Merci. Alors c'est un amendement qui va évidemment dans le bon sens, car cela va permettre de faire face à la haute intensité en augmentant le nombre des équipes chirurgicales projetables et en étudiant permettant d'étudier les moyens de renforcer la médecine de l'avant en s'appuyant sur les compétences des infirmiers désarmés avis très favorable. Monsieur le Ministre. Je ne suis pas contre. Sur le fond, après on a déjà introduit par voie d'amendements successifs, l'équivalent d'une page entière dans le rapport annexé, service de santé des armées. Donc moi je m'en remets la à la sagesse. Enfin il y a pas de contresens dans ce que vous. Vous écrivez après je le renvoie à la réflexion globale de forme du rapport annexé donc de ce point de vue sagesse. Alors, avis favorable de la commission et sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons au 183 monsieur compte de madame Vogel donc Monsieur Salmon. Merci madame la présidente. Avant toute chose, je tiens à saluer l'engagement pris par le gouvernement qui promet par cette loi de programmation de moderniser le ravitaillement médical notamment ses capacités de stockage et de production dans le contexte des pénuries de médicaments, c'est une mesure de bon sens, une mesure inévitables cependant nous repris regrettant que cette disposition laisse une marche une large marge de manoeuvre pour ne pas dire qu'elle est floue. Pour y remédier. Nous proposons d'y apporter 3 précisions, premièrement, nous souhaitons que les stocks de matériel médical et de médicaments soient considérablement augmenté. Deuxièmement, nous souhaitons spécifié qu'il faut également stocker des médicaments pris sur une base régulière. Il peut s'agir d'antihistaminiques ou encore de médicaments anti-rétro-viraux. Il s'agit dès lors de s'assurer que ces personnes qui peuvent vivre sans complications avec le virus ait accès aux médicaments qu'il qu'elle prennent en général une à 2 fois par jour. Troisièmement, il faut préciser que les médicaments peuvent bien évidemment être administré aux militaires mais qu'il pourrait également être distribuées aux populations touchées par un conflit armé ou une catastrophe naturelle. Nous pensons que cette précision est essentielle et permettrait à l'armée de répondre en urgence à des besoins humanitaires. Nos forces armées ont l'infrastructure pour acheminer rapidement du matériel comme des médicaments dans des zones de crise. Il s'agit de mobiliser cette capacité pour venir en aide à des populations civiles qui ont tout perdu, là aussi, il s'agit non seulement distribuer de la pénicilline mais de penser aux personnes qui ont besoin d'un traitement régulier, merci. Quel est l'avis de la commission favorable au gouvernement défavorable je avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui compte qui s'abstient. Il est adopté le 115 messieurs Cigolotti. Oui merci ben à la présidente. Juste pour évoquer, toujours dans le prolongement de des amendements de mes collègues. Perrin et et Gontard. Le service de santé des armées. Ce service de soutien et l'un des seuls parmi. L'ensemble de, de nos alliés à disposer de de savoir faire tout à fait spécifique et. Je crois que nous devons faire en sorte de conserver ses savoir-faire même les États-Unis, même parmi nos alliés les plus importants. Nous sommes les seuls. À bénéficier de de certaines capacités et compte tenu du du risque de conflit de haute intensité. Il nous apparaît important à travers cet amendement que l'on puisse apporter une sécurité pour nos militaires projetés notamment en opération extérieure pour leur assurer un un maximum de chances de survie que le le ça soit en capacité, hé bien de d'apporter les services nécessaires à nos militaires. Donc nous demandons par cet amendement que le ministère des Armées engage ne travaille pour répertorier et conserver les savoir-faire du service de soutien.

Merci Alain la présidente. Les épreuves de sélection organisées en vue de recruter des militaires sont essentiels à bonne composition de nos armées. Or il s'avère que souvent. Une fois les épreuves de sélection. Effectuée on passe à la vice-médical et malheureusement une fois la liste et effectué, on se rend compte qu'un certain nombre d'inaptitude donc l'idée, l'idée de cet amendement et que les prérequis modique les prérequis médicaux soient communiquées par le service de santé des armées, aux candidats à l'incorporation, avant que ne débutent les épreuves de sélection. C'est pour éviter peut-être qu'on ne fasse venir des outre-mer ou autre pour des sélections et qu'on les renvoie ensuite et que ou pour des ou pour des nationaux qui qui aurait, qui serait dans cette situation-là, pour éviter de perdre un temps inutile et n'est évidemment pas question de demander au OSS de réaliser ces visites d'aptitude mais de trouver un dispositif qui nous permet en tout cas d'être plus efficace et de coûter moins cher à un autre les prérequis globaux font déjà le médicaux font l'objet évidemment de publication, par un arrêté du ministre de l'en charge de la Défense à chaque fois le sujet c'est évidemment. L'adaptation c'est prérequis et aux candidats en l'espèce, donc bon sagesse après on vient alourdir encore un peu le rapport annexé au Touquet, il y a pas de problème sur la publicité des prérequis globaux

merci madame la présidente, le parc de logements, hébergement aux militaires et à leurs familles et dans un état critique, a souvent délabrées par Ouest-thermique. Vous avez entrepris depuis quelques temps une tout un processus pour réhabiliter ces logements et finalement notre amendement viennent vous encourager à continuer dans la bonne direction. Parce que je pense qu'il faut offrir effectivement comme vous je pense à des conditions normales de logement digne à nos militaires. Et en plus ça contribue à la fidélisation donc on vous a courage à continuer dans cette direction et on ajoute à cela la référence à la loi climat et résilience. Avis de la commission favorable avis du gouvernement. Sagesse dans le même esprit de ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur la forme du rapport annexe. OK. Qui est pour.

qui du coup interdit en 2028 le la location des passoires thermiques donc qui veut dire que en 2028 on ne pourra plus. Utiliser des logements s'ils n'ont pas été réhabilité. Moi ça me va très bien, mais du coup on m'avait, on avait fait le retour. En commission, avec un avis défavorable sur mon amendement en me disant que c'était très compliqué. Que si on ne tenait pas, on pouvait pas se permettent quand même de ne plus pouvoir. Utiliser ces logements pour les pour les troupes et c'est pour ça qu'on avait rédigé un amendement moins contraignant qui vient juste juste après. Qui permet de suivre cet objectif mais d'être beaucoup moins contraignant parce que effectivement ça peut être assez complexe en 2028 de ne plus pouvoir utiliser. Ces logements, s'il n'était pas rénové même si effectivement l'objectif c'est bien de les rénover le plus rapidement possible. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Oui je vous aviez tous retenus, qui avait un avis favorable de la commission de sagesse du gouvernement Monsieur Gontard le 229.

Mais ne vous éloignez pas Monsieur Gontard. Vous avez encore le 230 231 le 232 le 233, c'est Monsieur Salmon, qui les prend. Oui merci la la présidente on on se partage un petit peu le le plaisir donc. Cet amendement. C'est pour un audit pour demander des audits réguliers sur les bâtiments les installations militaires. Le mystère de la Défense et le ministère le plus énergivore de l'État français avec une consommation de 850.000 m3 de produits pèse pétroliers. Il apparaît donc nécessaire qu'ils fournissent des efforts importants en la matière, les audits énergétiques permet d'identifier les sources de gaspillage d'énergie les inefficacité énergétique dans les bâtiments les installations militaires afin d'y pallier et de réaliser des économies de coûts significatives à long terme. Poser un diagnostic général permettra de construire un plan global échelonner la rénovation du bâti militaire. Par ailleurs, au-delà du souci de limiter les coûts et l'impact environnemental. L'enjeu est hautement stratégique, il s'agit de réduire la dépendance des armées françaises aux approvisionnements en pétrole à l'heure où les tensions géopolitiques s'accroissent dans le domaine de l'énergie. Comme a pu l'expliquer Madame Parly les ressources sont de plus en plus localisés dans des zones de conflit ou au sein de pays qui n'hésite pas à l'utiliser à utiliser l'arme énergétique pour limiter notre liberté d'action, notamment la Russie ou les pays du Golfe et alors même que nos besoins augmentent. Par ailleurs il est encore une fois question du confort de nos militaires confrontés au problème des passoires énergétiques également merci. la rédaction qui est proposée, nous paraît inopportune dès lors que nous ne disposons pas d'une évaluation des coûts associés à l'organisation d'un audit énergétique de l'ensemble des bâtiments et installations militaires qui doivent bien évidemment rester cohérent avec la trajectoire budgétaire adopté par le Parlement. Je pense que nous on a un travail ultérieur pour évaluer les coûts et programmée cet audit. Et je vous propose de retirer cet amendement. Madame la Ministre même vie. Oui merci madame la impression la ministre. Monsieur le le député dès lors que cela ne limite pas ses activités opérationnelles coeur de sa mission. Le ministère des Armées porte une trajectoire ambitieuse de décarbonation de ces bâtiments, de développement de recours aux jets aux énergies renouvelables et de sobriété énergétique Attestent les différentes stratégies énergétiques du ministère sur le fond les emprises des bâtiments énergivores sont ciblés prioritairement et nous signalons la sous cette LPM. Pour un exemple concret, le remplacement de l'ensemble des chaudières de fioul est programmée selon les objectifs fixés pour leur suppression en 2031 des objectifs ambitions seront suivies dans le cadre de de la stratégie militaire, de la performance énergétique et d'exemplarité de 2022 et du plan Ambition logement et sur le second et Crémant du programme hébergement dans le cadre du plan de rénovation des ensembles d'alimentation et de loisirs voilà. Des efforts sont engagés depuis plus de 10 ans ont porté leurs fruits. La consommation énergétique totale du parc immobilier des armées a baissé de plus de 20% entre 2010 et 2023 dans le même temps les consommations d'énergies fossiles et les hommes et les émissions de gaz à effet de serre associés ont été. Diminué de près de 30%. À terme, l'objectif de réduction de consommation énergétique par rapport à 2010 et de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Enfin, compte tenu du Patrimoine immobilier opérationnel et tertiaire du MIN armes votre amendement demande un audit extrêmement lourd et coûteux pour le ministère, alors même qu'il est engagé sur la transition énergétique. Je vous propose un retrait. Monsieur le président Gontard pour une explication de vote. merci merci madame la présidente. Dans juste juste rappeler que le le dit extrêmement lourd, c'est celui qui est demandé à l'ensemble des personnes qui vendent par exemple lors lors bien donc c'est pas un audit de enfin voilà c'est ce qu'on demande à tout à chacun et, et deuxièmement, si on veut tenir l'objectif de l'amendement qui vient d'être voté pour une rénovation thermique de l'ensemble des enfin des bâtiments et de les sortir des passoires thermiques d'ici 2028 on aura besoin de faire ces audits énergétiques, donc en fait c'était plutôt un amendement de logique en fait. Et, et d'avoir justement cette cette obligation en tout cas de faire ces audits pour pouvoir détecter justement les bâtiments qui sont des passoires thermiques et ensuite pouvoir intervenir dessus, donc c'était plutôt un amendement vraiment de cohérence. Très bien, jamais aux voix donc double avis défavorable qui est pour.

et doivent passer par tous les pans de la société en ce sens, l'armée est également concernée elle doit contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de la France et pourquoi l'amendement que nous proposons demande qu'à chaque fois que c'est possible. Des dispositifs de production d'énergie solaire sont installés sur les toitures des bâtiments. Nous sommes bien conscients que l'installation de ces dispositifs peut représenter un coût initial élevé cependant ces investissements généreront à long terme des économies grâce à la révision des coûts de l'énergie. Les infrastructures militaires comme. Hangars sont particulièrement bien adapté à l'installation de ces dispositifs grâce à leurs grands espaces en plus un Avantage financier. L'installation de panneaux photovoltaïques présente un Avantage stratégique puisqu'elle permet à l'armée d'améliorer son autonomie énergétique en réduisant la dépendance aux sources d'énergie extérieure. L'armée est une institution publique. Par conséquent, elle se doit de montrer l'exemple dans tous les domaines et donc dans le domaine de la transition énergétique en augmentant son utilisation d'énergies renouvelables. L'armée enverrait un signal fort et positif à la société française et contribuerez et contribuerait à l'éducation et à la sensibilisation du public sur ces enjeux. Il s'agit ici de faire participer l'armée aux objectifs de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, ainsi que de commencer à appliquer les dispositions de la directive européenne sur les énergies renouvelables, adoptée le 16 juin dernier.

on partage le même objectif. Effectivement il y a bien sur le plan place au soleil, avec les 2000 hectares de terrain consacrés au développement de projets de production d'électricité photovoltaïque j'étais il y a pas longtemps en novembre à Arcueil. Où il y a eu un bâtiment justement pour les cadres qui a été inaugurée où on peut récupérer. Aussi. Sur le toit avec avec l'énergie solaire il y a sur la base de 125 à Istres 4 bâtiments qui sont en train d'être construit et qui aurait été évidemment réfléchi non pas. Uniquement sur sur les énergies renouvelables, mais aussi sur le positionnement des bâtiments pour faire en sorte que, avec les vents, ils puissent avoir moins de dépense d'énergie. Alors sur le fond, je vais vous donner un avis de sagesse parce que et c'est parfois c'est mieux de l'écrire.

Merci madame la présidente, c'est bientôt. Terminé comme nous l'avons déjà rappelé à plusieurs reprises la transition énergétique par passe par des efforts collectifs qui doivent se mener au sein de tous les secteurs de la société et de l'armée en fait évidemment partie. Et en ce sens nous avons choisi de proposer un amendement qui vise dans le même sens que celui qui vient de que je viens de décrire qui vise à envisager le déploiement d'éoliennes sur les emprises militaires au même titre que l'installation de panneaux solaires, l'installation d'éoliennes représentera sans aucun doute un coût initial élevé elle permettra à long terme une baisse du coût de l'énergie importante en effet, le ministère de la Défense dispose de plus de 250.000 hectares d'emprise qui n'accueille à ce jour pas ou peu d'éolienne, la possibilité de déployer des éoliennes sur les emprises militaires avaient été envisagées par le gouvernement pendant les travaux préparatoires de la loi sur le développement des énergies renouvelables. Il a depuis renoncé à cette possibilité, sans que l'explication ne soit parvenu. Pourquoi ce renoncement à quelles conditions. Ce déploiement est-il possible et de quelle marge de progression disposerons-nous quels obstacles existe-t-il encore pour envisager de déployer des hooligans sur les emprises militaires qui demeure l'un des rares gisements possible de développement de l'éolien terrestre en France. sur cet amendement, la Commission constate que nous n'avons aucune étude de faisabilité de ses installations. Ni une ni aucune évaluation des coûts associés. Un travail ultérieur permettra d'aller certainement plus loin à défaut c'est soit un retrait soit un avis défavorable. Avis du gouvernement. Oui alors vous avez vous avez mentionné le fait de pas avoir eu d'explication sur. Sur. Les intentions du gouvernement Pour vous dire sur les emprises militaires. Ça pose un souci c'est que les éoliennes pour un grand nombre de raisons ne peuvent pas être positionné sur les emprises militaires pourquoi. D'abord parce que les éoliennes performante. De grande taille sont des obstacles. À l'envol et à la circulation aérienne. Elles ne peuvent donc pas être installés sur les bases aériennes ensuite toute emprise. Il y a un radar de brouillage ne peut, ne peut pas accueillir aussi d'éoliennes et puis pour la 3ème raison toute emprise ayant une zone de largage ne peut pas accueillir non plus d'éoliennes.

Madame la Ministre la réglementation environnementale 2020 s'applique déjà aux logements bureaux ainsi que tout bâtiment militaire faisant l'objet d'un permis de construire. L'amendement que nous proposons vise simplement élargir autant que possible les préconisations essentiel de la 20 20 aux autres constructions militaires. L'objectif de cette réglementation et de poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions tout en diminuant leur impact carbone et le permet des constructions durables autosuffisante en énergie construites en matériaux biosourcés s'appuyer sur nos filières locales et favoriser la fin de vie, la moins impactante des bâtiments le. Domaine de du militaire n'est pas hors société et donc doit s'emparer complètement de la question de la transition écologique comme pour le reste. Oui madame la présidente. Cet amendement vise à. À lutter conte la frilosité des des secteurs bancaire et financier de financer les industries de défense en raison des risques tout en conformité juridique et réputationnel. Il est nécessaire de faciliter l'intégration de la BITD dans le Champ de financement de ces mêmes institutions. L'augmentation du coût de financement engendre un désavantage de notre BITD, comme nous avons pu le constater en de maintes occasions vis-à-vis notamment des compétiteurs. Non. La réduction de la capitalisation boursière des entreprises quant à elles du secteur pose également un risque de prise de contrôle par les investisseurs étrangers. Avis de la commission. Oui. Face à la frilosité de la part de certains établissements bancaires et des d'établissements financiers. Cet amendement va dans le bon sens. Donc il faut aider ces établissements à prendre leur part dans le soutien à la BITD, un avis favorable. Monsieur le Ministre oui sagesse. Et ce temps avis favorable de la commission avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Monsieur tu es mal le 92 ans. Il est défendu. Quel est l'avis de la commission. Favorable Favorable avis du gouvernement défavorable. Défavorable je mais on voit qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Nous avons. Monsieur de Lège le 125. Merci madame la présidente. Il s'agit de reconduire dans l'actuel. 1er Damasio militaire. Un dispositif qui existait dans l'ancien et qui stipule que en cas de cession. Eh bien le prix de cette session revient au ministère. Avis de la commission favorable avis du Gouvernement. Sagesse mais favorable. Alors sur cet amendement favorable de la de la commission sagesse bienveillante du gouvernement qui est pour. qui s'abstient. Il est adopté un amendement du gouvernement maintenant le de 79. Il est défendu avec les mêmes arguments que précédemment. Madame la présidente. Merci à l'avis de la commission. Favorable Favorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Monsieur Perrin. Le 64. Mais. Ailleurs, pardon, excusez-moi. L'amendement de notre collègue Perrin met l'accent sur le rôle des PME et ETI dans le processus d'innovation. Les PME et ETI innovante hésite en effet parfois à se lancer sur les marchés. Faute de président. Prévisibilité. Des commandes et de financement suffisant pour initier des projets les moyens consacrés aux études doivent permettre d'accompagner ces structures afin de favoriser leur croissance et stimuler l'innovation dans le tissu industriel puis envisager une enveloppe à hauteur de 10%, soit environ un budget de 100 millions d'euros par an. Avis de la commission favorable avis du gouvernement. Oui ce geste. Alors ai mis aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Madame Carlotti 93. Défendu avis de la commission demande de retrait, retrait. Monsieur le Ministre votre donc double avis défavorable. Voilà. Vous vous voulez faire une explication de vote peut être. Oui parce que oui parce que nous avons voté exactement la même chose dans le corps du texte.

le rapport annexé avec le texte de la loi. Donc voilà je sais qu'il y avait une opposition du gouvernement sur ce point, pas de la commission à l'époque. Eh bien je vais quand même le métro voix et qui est pour. Et qui est contre et qui s'abstient et il n'est pas adopté et maintenant le 315 du gouvernement. Oui madame la présidente, pardon pour le dépôt tardif mais il est le corollaire. Des amendements précédents de suppression qui est un engagement du gouvernement, donc vous pouvez prendre connaissance il est défendu naturel. Avis de la commission. Avis favorable car il répond au besoin d'information que le Parlement a exprimé sur tous ces sujets essentiels qui doivent nous conduire vers la préparation à la haute intensité.

Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Il comprend bien le sens de cet amendement. Mais ce n'est pas ce n'est pas le le rapport annexé n'est pas le véhicule adapté pour prendre des dispositions normatives sur la composition de la future commission il reviendra donc aux parlementaires en en fonction en 2028, de juger si les dispositions du gouvernement sont pertinentes. Donc, avis défavorable. Merci la vie de monsieur le ministre. Oui mais ma vie même argumentaire. OK. Retrait merci 2 amendements en discussion commune le 147. Monsieur le président. Il est retiré. Merci.

Avis favorable donc je mets aux voix l'amendement monsieur tu es mal pour. Explications de vote. Oui bien sûr. Non parce que je, je souhaite le le dire pour rendre hommage à monsieur Gilbert Roger qui a proposé effectivement cette cette idée de d'étude de la faisabilité de faire poursuivre encore quelques années le Charles-de-Gaulle. Il y a eu un amendement qui a permis d'atterrir et donc je souhaitais juste souligner qu'on avait pu avancer collectivement Gilbert Roger. La commission et bien sûr le gouvernement. Merci. Alors je vais donc mettre aux voix l'amendement 312 du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est donc adopté, je me vois l'article 2 qui est pour. Contre qui s'abstient. Il est donc adopté. Et maintenant je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des explications de vote.

puisque c'est vrai qu'on, on a commencé, souvent par les moins financier et assez peu par les éléments stratégiques mais c'est lié au fait qu'on n'a pas eu ce débat préalable et c'est pour cela que je souhaitais pas la parole. Dire que je crois que le le Sénat et je veux aussi remercier la la commission. Son président, l'ensemble des rapporteurs. On a su je crois collectivement. Et sensiblement le texte même si encore debout et je forme le voeu que nous puissions atterrir ensuite en commission mixte paritaire parce que je crois que c'est l'intérêt collectif et j'appelle le gouvernement à faire quelques bouger aussi pendant la commission mixte paritaire afin qu'on puisse élaborer et voter un texte commun. Je crois nécessaire pour nos armées. Merci. Alors Monsieur Cigolotti. Merci madame la présidente, monsieur mal là il y a ouvert les hostilités. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous voici donc arrivé au terme de l'examen de cette loi de programmation militaire pour la période 2024 2030. Pour notre groupe, nous ne pouvons que nous réjouir des apports du Sénat dans ce texte, oh combien structurants pour nos forces armées. Ce texte était attendu par notre commission bien sûr mais également par le militaire. Cette augmentation significative du budget de la nation consacrée à nos armées est la bienvenue. Monsieur le Ministre. Après des années d'érosion. Cette LPM poursuit le mouvement engagé dès 2019 et accroît l'effort financier nécessaire après le retour de la guerre sur le front oriental de l'Europe. Nous ne pouvons que saluer les efforts consentis pour nos différentes composantes. Bien sûr pour nos services de renseignement en y intégrant et c'est la vie de notre groupe. Le programme dédié au porte-. Avions de. De nouvelle génération. Même si nous avons eu quelques difficultés de compréhension, dûes à la différence d'affichage que nous avons désormais parfaitement intégré nous. Apprécions. Les accords qui ont été réalisés il appartiendra désormais à la CMP, c'est ce que vient d'évoquer notre collègue Rachid Temal de régler les quelques différends laissés en suspens et en tout cas, c'est la volonté de notre groupe, de pouvoir aboutir pour que cette loi de programmation militaire soit promulguée le plus rapidement possible. Merci à nos. Z'orateur merci à notre président rapporteur et merci à Monsieur le Ministre qui parfois a été long mais a été très pédagogue. Monsieur Lisa. Oui madame la présidente merci, juste quelques mots. Pour quand même noter tout le travail réalisé par la Commission, par son président, par les membres de la commission et et l'ensemble des administrateurs, on a quand même commencé ce travail au mois de novembre dernier. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des difficultés remercier aussi monsieur le ministre, on a eu parfois des échanges. Serrés technique mais à chaque fois on a eu des réponses et l'essentiel c'est de pouvoir aboutir et je crois, Monsieur le Ministre, j'ai le sentiment que vous repartirez du Sénat avec un texte finalement assez équilibré et peut être quelques prescriptions, on verra ce qu'il en sera à à la CMP mais mais je crois que vraiment il y a eu un travail extrêmement positif. Un travail de qualité fait et je voudrais remercier aussi. Certainement au nom des commissaires et l'air mais peut être aussi de l'ensemble des collègues. Le président Christian Cambon sur sa façon de travailler sur la façon dont il nous a fait travailler et je crois que si on a un résultat positif. Aujourd'hui c'est essentiellement dû à sa méthode, on a pu additionner nos forces à chaque fois que c'était nécessaire assumer nos différences et en parler quand il en avait et je crois que c'est un peu l'honneur du travail parlementaire. Merci monsieur le président Gontard. merci madame la la présidente. Après 3 jours de débats riches et intenses, nous nous nous demeurons cependant assez perplexe puisque vous refusez toute nouvelle recette, nous ne savons toujours pas comment sera financée cette ambitieuse programmation militaire et quel autre politique publique. Elle laissera cet angle mort nous empêche de voter en connaissance de cause. Ce que nous avons pu retenir en tout cas compris de nos échanges, c'est qu'en refusant de faire des choix en conservant modèle d'armée global en ni d'équations avec la réalité de notre puissance et de nos moyens en investissant tant sur la dissuasion nucléaire en multipliant les nouveaux espaces de conflictualité. Nous nous retrouvons, face à un double risque. Les temps si l'échantillonnage de notre armée où l'explosion colossale des dépenses des prochaine LPM pour continuer à financer tous ces nouveaux programmes très onéreux. Tout cela sans investir suffisamment sur les moyens humains et capacitaire notre armée de terre pour citer le poète la grenouille veut se faire plus grosse que le boeuf. Nous ne pouvons pas accepter un modèle d'armée qui oblige la France à refuser tout effort de désarmement nucléaire multilatéral un modèle d'armée qui repose sur la nécessité pour nos industriels d'exporter des armes sans aucun regard pour le respect des droits humains ou du droit tout court. Nous sommes convaincus que le modèle d'armée française doit être rationalisée et intégré dans une perspective de coalition européenne, même si nous n'ignorons pas qu'à court terme au moins cette Europe de la défense aura autant pour cadres de structuration. L'Europe et l'échelle pour retrouver la puissance à laquelle la France inspire pour faire face aux nouvelles menaces comme pour mutualiser nos efforts, nous avons trop de défis à relever pour laisser filer indéfiniment nos dépenses de défense. Nous souhaitons d'ailleurs que le gouvernement soit aussi réactif et ambitieux pour assurer notre sécurité climatique que pour assurer notre sécurité militaire cependant considérant l'urgente nécessité de reconstituer nos stocks pour continuer à aider l'Ukraine et considérant les progrès du texte enregistré au Sénat. Les écologistes dans leur très grande majorité s'abstiendront sur ce projet de LPM. Merci monsieur le président, Laurent. Merci madame la présidente. D'abord je voudrais remercier le président. Quand bon pour. Le climat de travail dans dans la commission, même quand nous n'étions pas d'accord. Remercié le ministre aussi pour les réponses directes qui l'a fait aux différents arguments qui étaient. Présentés tout au long du du débat. Nous allons voter contre cette loi de programmation. Qui reste à nos yeux, marqués par un défaut de conception stratégique une analyse simpliste des causes de la conflictualité. Cette. Loi de programmation en douce. Une augmentation très forte des dépenses militaires évidemment mais. Tout cela dans un. Dans un climat général de réarmement mondial qui est précisément une des causes de la montée des conflictualités et qui n'est pas une solution. Assez conflictualité. Nous pensons nous-mêmes qu'il y a besoin d'augmenter les dépenses dans un certain nombre de domaines, dont l'équipement de nos forces dans le maintien en condition opérationnelle dans un certain nombre de domaines les drone par exemple. Mais dans d'autres. Nous avons beaucoup de de doute pour pas dire plus, et je les ai exprimées ici. Sur plusieurs domaines où nous accompagnons une militarisation grandissante qui je crois est inquiétante. La LPM est adossée à une stratégie d'engagement totalement imbriquée à celle de l'OTAN. D'ailleurs le débat, je trouve très éclairant que nous avons eu sur les raisons pour lesquelles il fallait à tout prix maintenir. L'objectif des 2%. Quelle que soit sa. Sa validité budgétaire je dirais a été très éclairant de ce point de vue, on a bien compris qu'il s'agissait d'un affichage politique de notre implication. dans l'organisation. De l'Alliance Atlantique. Et. Nous le faisons je crois au détriment de, de la recherche d'alliances stratégiques ouverte qui préserverait davantage notre indépendance dans ce monde mouvant la LPM met à l'écart, la prévention des conflits tout objectif de désarmement. Je conclus. Et sur le nucléaire. Elle passe à côté de la réouverture d'une réflexion plus globale en refusant notamment que nous participions comme membre observateur aux conférences du tuant voilà pourquoi très vit très rapidement résumé, nous voterons contre cette loi de programmation militaire. Merci monsieur. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président, rapporteur. Mes chers collègues. Tout d'abord le groupe RDPI partage les objectifs de cette loi de programmation militaire telle que présentée par le gouvernement. Elle permet en effet de donner à nos armées, des moyens à la hauteur des menaces. Protéiformes qui se profile. Depuis 5 ans déjà, le président de la République a engagé la réparation de nos armées après des décennies de baisses budgétaires la LPM 2019 2025, je le rappelle, a été exécuté à l'euro près. Une première depuis 40 ans. Ces effets concrets commence à se voir dans les régiments et dans les bases en France comme sur les théâtres d'opérations projetées. Demain la LPM 2024 2030 permettra d'amplifier cet effort afin de faire face aux menaces qui s'additionnent. Au total, le budget des armées qui était de 32 milliards en 2017 sera concrètement de 56 milliards en 2027 et de 69 milliards en 2030. en 2030. Il aura donc plus que doublé, sous l'impulsion du président de la République et l'ex-étant l'excellente déclinaison qui a pu en faire, le ministre des armées, aux côtés du Parlement. Cette hausse permettra notamment de moderniser notre dissuasion nucléaire d'investir massivement dans les nouveaux champs de conflictualité l'espace le cyber ou encore les fonds marins d'améliorer nos moyens dans les territoires d'outre-mer à hauteur de 13 milliards de doubler les effectifs de nos différentes réserves et de doter nos forces de capacité adaptée aux menaces et complète grâce à un effort de cohérence sur les munitions et sur le maintien en condition opérationnelle. Toutefois, certains amendements adoptés par le Sénat ont conduit à éloigner le texte de sa cohérence initiale. À ce titre, notre groupe s'interrogent sur l'impact budgétaire que pourra avoir l'ajout de plusieurs matériels supplémentaires. Et sans que soit mis en face les infrastructures et les soutiens les munitions et la formation qui vont avec. Aussi, cette version fait peser certaines contraintes nouvelles sur les acteurs de notre défense. En bref, les 2 lois de programmation militaire, décidée par le président de la République permettront de doubler le budget des armées. En cohérence notre groupe votera pour ce texte, dont l'ambition sans précédent depuis des années 60 n'a pas été dénaturé. À l'issue de nos débats. Merci. Merci madame la présidente, de nous venant d'examiner, dans un esprit globalement de sagesse. Un projet de loi de programmation militaire dont le montant colossal. J'ai dit bien colossal de 413 milliards d'euros est à la hauteur des défis. La France a besoin de son armée, une armée performante capacité de faire face aux nouvelles menaces et de répondre à ses engagements internationaux, tant au niveau européen. À l'issue de la lecture du test par le Sénat, nous pouvons nous satisfaire de certaines dispositions, en particulier celle adoptée dès le stade de la commission, je pense à la révision de. La trajectoire budgétaire et la sécurisation des ressources ainsi qu'aux mesures de soutien à notre industrie Je n'oublie pas bien sûr aussi des améliorations concernant l'actualisation de la LPM qui permettront d'associer au bon moment et plus directement le Parlement pour les choix. Majeurs qui engagent notre outil de défense derrière les grands équilibres budgétaires, il y a bien sûr des hommes et des femmes qui font l'honneur de notre pays par leur engagement d'hier et d'aujourd'hui. Quant aux militaires d'aujourd'hui et ceux qui s'engagent à travers la réserve ou un apprentissage militaire pour les plus jeunes, ils se voient confortés dans leur choix par une politique d'attractivité et de fidélisation plutôt volontaire. Mais, chers collègues. Au-delà des désaccords que l'on peut avoir ici et là sur certains volets du test, le consensus républicain guide bien souvent le vote des crédits de l'armée. Le groupe RDSE prendra une nouvelle fois ses responsabilités en votant le projet de loi de programmation militaire 2024 2030 merci. Merci. Alors Monsieur le Président Cambon. madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre chers collègues nous arrivons donc ainsi au terme de nos débats sur un texte particulièrement important. La densité de nos échanges. La conviction qu'il a animé tous les sénateurs et les membres du gouvernement au cours de ces débats témoigne manifestement de l'importance de ce sujet. Ce travail. C'est d'abord pour nous tous et toutes. Une façon de rendre hommage à cet instant, aux femmes et aux hommes de nos forces armées qui expose. Au quotidien leur vie pour la défense de la France et pour la paix. Je sais pouvoir parler au nom de tous nos collègues pour saluer leur engagement et leur exprimer notre soutien et notre reconnaissance. Nous avons bien sûr également une pensée pour le lot blessés et pour ceux qui malheureusement ont donné leur vie pour la France. Depuis le vote de la dernière LPM en 2018 ainsi qu'une pensée particulière pour leur famille. Sur le fond. Chers collègues, nous avons tous souligné évidemment l'importance de l'effort budgétaire qui a été consenti pour les années 2024 2030. Dans un monde toujours plus instable toujours plus dangereux. Il était indispensable de poursuivre le redressement de notre effort de défense qui fait suite à plus de 20 ans des. Nous donnons acte bien volontiers. Monsieur le Ministre tente au président de la République qu'au gouvernement pour. S'être engagé dans cette voie du redressement. Alors bien sûr nos débats ont donné lieu à quelques divergences d'analyse avec le gouvernement en vérité sur grand de grandes catégories de sujet, le sujet de la programmation militaire avec peut-être cette ambiguïté qui a qui a créé le fait de discuter d'une enveloppe de programmation au lieu de discuter d'une enveloppe de crédits les parlementaires ayant plus l'habitude de discuter de crédit et aussi donc ceci a entraîné un certain nombre de divergences concernant les contours de l'exacte. Ambition capacitaire porté sur ce texte. Mais les échanges ont été francs et à l'heure qu'il est le dialogue a été ouvert et je suis plus que jamais persuadé que nous allons arriver à. Obtenir un accord et nous allons converger tant avec le gouvernement qu'avec nos collègues députés de la de la commission mixte paritaire qui va se tenir le jeudi 6 juillet. Le second axe sur lequel nous avons évoqué nos bien des sujets c'est le contrôle par le gouvernement de l'exécution de ce texte, c'est une conviction profonde du Sénat, vu les sommes en jeu, il est indispensable que le Parlement participe au portage politique de cet effort de défense. Monsieur le Ministre de la robustesse et la crédibilité de la LPM en dépendent véritablement permettez-moi enfin de remercier bien sûr les différents présidente et président de séance qui ont permis la meilleure tenue de nos débats. Je veux remercier bien sûr tous les orateurs des différents groupes au-delà de nos différences légitimes de sensibilités politiques, nous avons défendu nos points de vue dans un esprit de respect et d'écoute et je suis fier d'avoir permis à chacune et à chaque groupe qui constitue notre commission d'avoir pu participer de manière concrète par l'adoption d'un certain nombre d'amendements à la à l'édification de ce texte. Monsieur le Ministre, nous on nous échangeons parfois été tonique c'était un plaisir avec vous. On a eu des des des divergences et c'est bien normal. Le rôle du Parlement, on le sait et vous le savez mieux que tout puisque vous appartenez quelque part à cette maison. Le rôle du Parlement c'est d'analyser de critiquer lorsque c'est c'est nécessaire et aussi de je souhaite saluer à cet instant, votre engagement personnel dans la très lourde mission qui est la vôtre et votre dynamisme et je salue bien évidemment les ministres et des secrétaires d'État qui vous ont entouré et accompagnés tout au long de cette mission. particulièrement avec un soin. Tout particulier. Les rapporteurs. Qui monte. Aidez-les 8 rapporteur qui m'ont aidé dans ce travail, ça a été un travail très long. Mais véritablement, qui a été fait dans un esprit. De recherche systématique de l'intérêt supérieur de notre pays et je veux véritablement leur dire ma fierté d'avoir pu conduire ses travaux avec chacune et chacun d'entre vous, avec vos sensibilités respectives. Alors nous allons dans quelques instants. Achevé ce travail parlementaire qui co-se conclura, dans le cas de la CMP. Je conclus en vous disant comme j'avais dit il y a 5 ans à votre prédécesseur et des-nous à vous aider et donc le dialogue qui a été engagé va certainement nous permettre de donner à nos armées, une programmation forte, une programmation robuste à la hauteur des enjeux. Enfin, d'un mot personnel. Je veux vous dire que ce fut un, c'est un honneur et ce fut un honneur pour moi. De rapporter cette 2ème LPM puisque j'avais eu l'honneur aussi de rapporter la première, je pense que je n'aurais pas le plaisir de de rapporter la troisième mais en tous les cas ça a été pour moi un moment tout à fait important et je veux donc partager avec vous toutes et tous, le sentiment d'avoir oeuvré au renforcement de nos armées qui reste pour moi et pour nous tous, la meilleure garantie pour la sécurité et la souveraineté de notre de notre pays. Merci à tous. Alors je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense j'ai été saisi d'une demande de scrutin public à par la Commission et par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Alors résultat du scrutin. Nombre de votants 343 exprimés, 331 pour 314 contredisent tête le Sénat a adopté. Et je vais donner la parole tout de suite à monsieur le ministre. Je la réclamais pas madame la présidente, le Sénat a adopté le Sénat s'est exprimé. Merci pour les débats. J'ai la, j'ai la faiblesse de penser que. Les sujets de défense et de sécurité collective, ce sont des sujets éminemment politique et techniques mais avant tout éminemment politique 2ème conviction notre constitution. Hé bien fait et le rôle de chacun, du président de la République du gouvernement mais aussi du Parlement a été bougrement bien imaginé par Michel Debré, entre autres. Et notamment dans le dialogue qu'il a eu avec. Les partis de gauche, issue de la 4ème République aisance là les mémoires de Michel Debré. Les travaux qui ont été conduits sur le rôle la relation qu'il avait avec la défense nationale était intéressant et je trouve que les, les débats ont permis de le faire trois le président comme on l'a dit 2 thèmes ont fait l'objet d'une grande discussion le contrôle ou. Comment le Parlement est éclairé et les manières dont il peut évidemment exercer ses missions constitutionnelles sur une loi de programme ont fait l'objet de de débats intéressants et je crois d'avancer, je pense qu'il y aura un calage encore en tout le CNL et l'Assemblée nationale je des sujets au fond d'ailleurs qui ne sont pas des sujets si lourd que ça, pour le gouvernement mais je pense que au nom du bicamérisme plus s'est exprimé clairement par le pouvoir législatif que ces consensuel les revoyure et mieux ce sera et puis évidemment. Un éléphant majeur dans la pièce et dans l'hémicycle à à à levé à soulever et à contourner, c'est évidemment une programmation budgétaire désormais qui va au-delà de la somme que le gouvernement avait initialement prévu et qui donc nécessairement devra amener une discussion. Entre les deux chambres et peut être avec le gouvernement pour faire en sorte de faire rentrer l'oreiller dans l'édredon puisque les engagements politiques qui ont été pris par les uns et les autres étant de ne pas dépasser les 413 milliards. Il reste donc un travail important à faire, je partage l'optimisme du président Cambon puisque à certains égards, effectivement j'ai été élu dans cette maison, donc je tâcherai de là où je suis comme membre du gouvernement aujourd'hui de la compagnie. Merci à tous. Merci, monsieur le Ministre. Alors, mes chers collègues, je vais lever la dernière séance de la session ordinaire. À partir du lundi 3 juillet le parlement sera réuni en session extraordinaire. Prochaine séance lundi 3 juillet à 16h pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à donner à la douane, les moyens de faire face aux nouvelles menaces et la séance est levée.